La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 31 janvier 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté.

La force du système français des brevets découle principalement de son intégration dans le système européen des brevets. Il y a une quarantaine d'années, la France a fait le choix, de sous-traiter à l'Office européen des brevets, l'OEB, la recherche d'antériorité. Les déposants français disposent ainsi d'un rapport de recherche, c'est-à-dire de nouveauté- est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? -, d'une très grande qualité, auquel est annexé un avis sur la brevetabilité- nous en parlerons tout à l'heure -, qui porte non seulement sur la nouveauté, mais aussi sur l'activité inventive. Disponible en moyenne neuf mois après le dépôt,

une grande organisation qui s'appelait l'Institut international des brevets, qui se trouvait à La Haye et que la France avait créée avec quelques autres pays. En plus, lorsqu'ils décident de procéder à une extension européenne de leur brevet dans un délai de douze mois à compter du premier dépôt, les déposants français bénéficient d'une réduction significative de la taxe de recherche et peuvent sans délai demander à l'OEB de procéder à un examen complet. Dans certains cas, le brevet européen est même délivré directement sans discussion ni modification de la demande. Il convient de préciser que le taux d'extension des demandes françaises par l'OEB s'élève à environ 75 %, contre 45 % en moyenne pour les autres pays. Cela prouve que les brevets français sont suffisamment solides pour mériter d'être déposés à l'étranger. Enfin, la force du système français des brevets est confirmée par l'analyse des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris, qui a une compétence exclusive en matière de brevet : le taux d'annulation des brevets français s'élève à environ 20 %, alors que celui des brevets d'autres pays est proche de 40 %. Je voulais rappeler ces éléments pour que nous ayons bien en tête le fait que le brevet français est un titre fort.

l'innovation est devenue une condition du développement de nos entreprises. Si les pouvoirs publics ne peuvent pas innover à leur place, ils peuvent leur offrir un environnement juridique propice à cette innovation. C'est l'objectif recherché par le présent projet de loi au travers du renforcement de la protection des titres de propriété de nos entreprises, et en particulier- j'insiste -des plus petites d'entre elles. L'innovation a un coût non négligeable. Les entreprises sont donc d'autant plus enclines à investir dans l'innovation qu'elles savent que celle-ci ne pourra pas leur être volée facilement par un concurrent et qu'elle valorisera durablement leur capital immatériel. C'est ce que permet le texte que nous examinons aujourd'hui au travers de deux mesures. D'abord, l'article 42 permet aux entreprises de contester plus facilement un brevet avec l'instauration d'une procédure administrative d'opposition aux brevets. Jusqu'à présent, seule la voie judiciaire était à la disposition des entreprises, ce qui dissuadait les plus petites de défendre leurs brevets, souvent faute de moyens, et les poussait à accepter des conditions défavorables à l'issue de transactions avec leurs concurrentes ou avec certains de leurs partenaires commerciaux. Ensuite, l'article 42 permet à l'INPI de s'assurer que les conditions de brevetabilité d'une invention sont réunies avant d'accorder le brevet. nous étions dans une situation paradoxale, dans laquelle la loi fixait les critères auxquels doit obéir tout brevet, mais les entreprises n'étaient pas obligées de les respecter et l'INPI ne pouvait pas s'y opposer. L'article 42 met un terme à cette exception française, qui affaiblissait non seulement la qualité des brevets français, mais également leur notoriété sur le plan le plan européen et mondial. Alors, non, cet article n'a pas vocation à affaiblir le brevet français au profit du brevet européen. Au contraire, il le rend plus compétitif, en améliorant sa qualité, tout en garantissant un prix d'accès toujours

À titre personnel, je fais confiance à notre rapporteur, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui défend le vote des dispositions proposées par le projet de loi sur les brevets. L'amendement

: protéger les créateurs et inventeurs, sans que cela entre dans le champ de la privatisation totale afin de préserver l'intérêt général. Mais il y a une réalité intangible : l'équilibre se rompt année après année, réforme après réforme, pour tendre vers une privatisation des inventions et des créations. Cela est allé tellement loin que la jurisprudence a dû elle-même rappeler que le droit de la propriété ne pouvait se placer au-dessus des droits fondamentaux. Alors, oui, on peut comprendre que les inventeurs puissent jouir de l'exclusivité de leur invention durant les premières années de sa création. Cela vise tout à la fois à leur permettre de rentabiliser cette invention et à continuer de travailler dessus pour l'améliorer, sans que la concurrence joue à plein. Mais les pratiques régulières de certains industriels et groupes d'intérêts, notamment en matière de brevets et de licences, dépassent largement ce cadre. Nous pensons bien évidemment à l'industrie pharmaceutique, qui a fait l'objet de diverses études, notamment en Belgique. Certains exemples sont édifiants : ainsi, l'ajout d'une vitamine a pu permettre l'émission d'une nouvelle demande de brevet et créer des marchés monopolistiques indus, ainsi que des rentes largement supérieures pour un produit aussi efficace. D'ailleurs, il faut rappeler que Médecins du monde, Médecins sans frontières et dix-sept autres organisations ont attaqué devant l'Office européen des brevets le brevet d'un médicament contre l'hépatite C ayant fait l'objet d'un nouveau brevet contestable. De fait, les trois alinéas que vise cet amendement tiennent parfaitement de cette logique de maintien dans le domaine privé. Pourtant, de l'aveu même du Gouvernement, les certificats d'utilité sont particulièrement adaptés aux inventions à cycle de vie court- on peut penser aux prototypes ou aux inventions de technologies, dont on sait qu'elles seront périmées quelques années après. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la mise en place d'un certificat limité à six ans, permettant notamment à des repreneurs de travailler sur des projets et prototypes abandonnés. Le certificat d'utilité est donc autant un outil de protection qu'un moyen de stimuler la recherche. Il présente aussi des avantages non négligeables pour les déposants, puisqu'il coûte moins cher et ne nécessite pas de rapport de recherche. Pour finir, presque -sa durée de vie, tout en facilitant la transition entre une demande de certificat d'utilité et une demande de brevet, revient à renforcer les mauvaises pratiques que je viens

Un certificat d'utilité se différencie d'un brevet, notamment par une durée de protection plus courte, une procédure d'examen plus légère, une délivrance plus rapide et un coût moins élevé. Près de quatre-vingt-dix pays étrangers disposent d'un titre de propriété intellectuelle pouvant s'apparenter au certificat d'utilité, notamment l'Allemagne et la modèle d'utilité ». Les règles de droit concernant le certificat d'utilité sont très variables d'un pays à l'autre. L'objectif de cet amendement est de rapprocher le certificat d'utilité français des modèles d'utilité allemand et chinois, chinois, qui ont déjà fait leurs preuves, en particulier sur leur champ d'application, leur système judiciaire et la possibilité d'un dépôt conjoint d'une demande de modèle d'utilité et d'une demande de brevet sur une même invention. Des mécanismes sophistiqués d'articulation ont été prévus dans ces pays, ne compliquant en aucune manière la procédure de dépôt. De tels instruments sont à prévoir et l'amendement vise donc à renvoyer à un décret en Conseil d'État le besoin de préciser les modalités techniques d'application.

effet, le brevet et le certificat d'invention n'ont pas vocation à protéger les mêmes inventions et il existe une progressivité dans la protection apportée par ces titres.

la France ne permet pas aux déposants d'une demande internationale d'entrer en procédure française, les privant ainsi de la possibilité d'obtenir un brevet français par cette voie. Elle les oblige de ce fait à s'adresser à l'Office européen des brevets. C'est seulement par un brevet européen qu'ils peuvent obtenir la protection de leur invention en France. Je rappelle que l'Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres, n'ont jamais opté pour une telle restriction dans leur propre droit. Les déposants du PCT peuvent ainsi demander un brevet directement auprès des offices allemand et britannique, confortant ainsi le rôle international de ces derniers. Il est proposé, cet amendement, d'abandonner cette restriction prévue à l'article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle, et ce pour plusieurs raisons. Il s'agit de permettre aux déposants internationaux d'obtenir un brevet français par la voie du du PCT et aux PME qui sont les utilisatrices types du système judiciaire français pour les litiges liés aux brevets de conserver cet avantage. Il s'agit aussi de maintenir économiquement les revenus liés aux litiges de brevets en France et de compenser l'impact sur les finances de l'INPI du futur brevet européen à effet unitaire. Enfin, cet abandon permettrait de conforter la procédure et les juridictions françaises compétentes en matière de brevets dans le futur contexte marqué par le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet. Cet amendement prévoit, la suppression de l'article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, afin de permettre à l'INPI de se préparer à jouer son rôle d'office de traitement direct des demandes internationales dans le cadre d'une phase nationale PCT.

Devant l'Assemblée nationale, la ministre chargée de la recherche a déclaré que cet article « était un élément fondamental de ce projet de loi ». Néanmoins, depuis vendredi dernier, le contexte politique de l'examen de cet article a radicalement changé. En effet, à l'occasion d'une grande réunion publique organisée pour célébrer les 80 ans du CNRS, le Premier ministre a lancé, de façon très solennelle, un grand débat national sur la science. Il le souhaite Il le souhaite le plus large et le plus libre possible et demande aux scientifiques de répondre à trois questions : « Comment garantir que les projets les plus novateurs soient financés au bon niveau ? Comment rester compétitifs à l'échelle internationale ? Comment convertir les découvertes scientifiques en innovations ?

Selon ce rapport, « l'incitation des chercheurs à se préoccuper de la valorisation est un enjeu essentiel. À cette fin, l'État a privilégié l'outil de l'intéressement et l'a rendu de plus en plus favorable au fil du temps. Néanmoins, Néanmoins, d'autres outils non financiers pourraient être mis en place pour lever les freins à l'implication des chercheurs publics dans la valorisation ». La démarche doit donc être plus systémique et il convient d'associer les chercheuses et les chercheurs à cette réflexion globale. C'est l'objet du grand débat national sur la science lancé par le Premier ministre. Je crains que les corrections que vous nous proposez d'apporter

et économique, repose sur notre capacité à investir dans les technologies de rupture. Si nous continuons à séparer et à cloisonner le monde de la recherche et celui de l'entreprise, notre économie ne réussira pas. Nous avons des concurrents asiatiques, par exemple chinois, et américains qui permettent aux chercheurs et aux entreprises de travailler main dans la main pour le plus grand bénéfice de ces nations. Je vous propose simplement de faire de même, en rehaussant la possibilité pour les chercheurs de passer plus de temps dans une entreprise.

Le statut de la fonction publique impose aux fonctionnaires des droits et des devoirs. Ces devoirs sont essentiels et permettent à l'État de disposer des compétences et du travail de ses fonctionnaires pour mener à bien ses missions au service de l'intérêt général, sous le contrôle du Parlement.

à Parme. Elle nous a expliqué que, à la suite des crises que vous connaissez- glyphosate ... -, elle avait été obligée d'écarter de son panel presque la moitié des scientifiques qui travaillaient pour l'agence en raison de leurs conflits d'intérêts. Elle demandait donc aux États membres, dont la France, de veiller à maintenir un corps de scientifiques qui en soit totalement préservé. C'est une nécessité absolue pour conserver la crédibilité scientifique et politique des avis rendus par les agences L'État en tant que tel, et non ses établissements, doit donc veiller, par le biais d'une commission de déontologie, à disposer d'une expertise scientifique totalement indépendante. C'est pourquoi nous proposons dans le présent amendement de rétablir les prérogatives

1 426 ont reçu un avis favorable, soit 91 % des cas. Il me semble important de faire confiance aux organismes de recherche qui connaissent bien les travaux de leurs chercheurs,

que j'estime supérieur. Si vous considérez que les avis de la commission de déontologie sont systématiquement favorables, je ne vois pas pourquoi ils constitueraient des freins

Je comprends parfaitement le raisonnement de M. le sénateur, qui souhaite permettre à un chercheur de participer plus activement à la gouvernance d'une société.

? Je m'en suis remis à la sagesse du Sénat sur l'amendement précédent, car j'estime que l'on doit pouvoir envisager que le chercheur ait une participation plus importante dans l'entreprise. En revanche, sur cet amendement, j'ai un avis clairement défavorable, parce qu'il pose un problème de principe.

qui nécessite un délai supérieur à un mois. Par ailleurs, vous souhaitez imposer un délai qui serait incompatible avec le droit de préemption des copropriétaires de l'invention.

En effet, les établissements publics de recherche concernés peuvent valoriser d'autres résultats de recherche que les inventions, par exemple, un logiciel, une obtention végétale ou un savoir-faire. La conclusion d'un règlement de copropriété, réglant notamment la répartition des droits de copropriété, est nécessaire pour procéder au dépôt et à la valorisation des résultats de la recherche. Cette information doit être portée à la connaissance du mandataire unique pour mener à bien ses missions, dans des délais compatibles avec la valorisation des inventions et leur exploitation par des industriels. Nous sommes bien dans le concret. bien dans le concret. Nous proposons que les dispositions qui seront prévues par voie réglementaire vaillent règlement de copropriété au sens de l'article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle, afin de permettre de déroger au régime de copropriété des brevets prévu par l'article L. 613-29 du même code, qui, lui, ne permet pas une valorisation efficace des brevets issus de la recherche publique. Ces dispositions pourront être complétées par convention.

en commission a conduit à ajouter aux critères objectifs de l'évaluation définis par le code de la recherche, aujourd'hui limités aux « contributions au développement de la culture scientifique et aux actions en faveur de la participation du public à la prospection,

De plus en plus nombreux sont mes collègues qui viennent exposer devant nos commissions leurs recherches sur des dossiers que nous traitons, et je m'en réjouis vivement, car nous avons collectivement beaucoup à apprendre de leur expertise. Parfois, les échanges que nous avons avec eux constituent de véritables innovations, parce qu'elles changent notre façon d'appréhender le monde. J'aimerais aussi que cet apport fondamental, plutôt d'ordre philosophique, politique, culturel, soit également reconnu dans leur carrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin,, je ne suis pas opposé à ce que les relations entre les chercheurs et le monde qui les entoure soient encouragées. Les dérogations consenties à leur statut sont peut-être nécessaires. J'aimerais alors comprendre pourquoi, quand il s'agit d'un parlementaire, il est indispensable d'établir une paroi totalement étanche entre sa carrière scientifique et son mandat. Je suis chercheur au CNRS en position de disponibilité pour la durée de mon mandat.

je vous rappelle que le code de la recherche dispose que « les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'entre elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

dans le cadre qu'a offert le Premier ministre aux chercheurs. Comme vous le dites très justement, madame la rapporteur, aujourd'hui, l'évaluation de chercheurs se fait en fonction de codes internationaux, mais qui ne sont pas du tout ceux que vous réclamez. Ils prennent

Contrairement à ce que disent les auteurs de l'amendement, ils autorisent des durées de recrutement plus longues et plus protectrices pour les salariés. Ils offrent en outre des garanties en matière de formation pour ces mêmes salariés. Par ailleurs, afin de prévenir les abus, il est prévu que la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier, ou une fois l'opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse. Pour conclure, je dirai que ces contrats offrent de nombreuses garanties aux salariés, tout en permettant de maîtriser la gestion du risque économique que font peser une activité et des financements par nature non pérennes dans le temps. L'avis est donc défavorable.

Par ailleurs, ayant moi-même commencé ma carrière professionnelle comme chercheur, attaché à la longue durée puisque je travaillais sur Marcel Proust, je reconnais bien volontiers la nécessité d'offrir du temps long aux chercheurs. Cependant, comme ministre de l'économie, je pense aussi que les Français sont impatients d'avoir des résultats dans le temps court. court. Ce projet de loi PACTE vise justement à concilier les deux : vous aurez le temps long pour le débat sur la recherche avec le Premier ministre, notamment sur cet établissement prestigieux, et qui fonctionne remarquablement bien, qu'est le CNRS ; pour ce qui est du temps court, je vous recommande de soutenir tout ce qui vise à faire tomber les murs entre la recherche et l'entreprise, ce qui nous permettra de créer des emplois tout de suite. Je pense que les Français sont impatients de les voir maintenant.

Cela fait des années que l'on entend ce discours sur la nécessité d'avoir des contrats courts, adossés à l'entreprise. À mon sens, ce qui fait le lien entre la recherche et l'entreprise,

propriété, condition tant pour encourager nos entreprises à innover que pour valoriser leur capital immatériel. Les dispositions qui nous sont proposées obéissent à trois objectifs adapter le niveau de protection ; renforcer la qualité des titres de propriété ; faciliter, notamment pour les PME, la défense de leurs titres de propriété en instaurant une procédure administrative d'opposition. Ces dispositions sont indispensables pour la compétitivité de nos entreprises. Or nous avons été nombreux à être interpellés avec insistance pour nous inviter à rejeter le dispositif proposé dans ce texte. C'est pourquoi, je souhaiterais revenir sur les arguments avancés par les opposants à cette réforme et mettre un terme à certaines contrevérités. On nous assure que le brevet français n'est pas si faible, puisque le taux d'annulation des brevets français serait inférieur à celui des brevets européens. C'est faux ! Depuis 2000, monsieur Yung, ce sont 41 % des brevets français qui sont annulés, contre seulement 23 % des brevets européens. Cela démontre donc qu'il y a un problème, lié à l'absence d'examen au fond des conditions de brevetabilité de l'invention par l'INPI. De même, on veut vous faire croire que ce fameux examen au fond découragera les entreprises françaises de se tourner vers le brevet national au profit du brevet européen, en raison de l'augmentation des délais et des coûts. Là encore, c'est faux Actuellement, le coût de la procédure devant l'Office européen des brevets, l'OEB, est de près de 5 000 euros, contre 636 euros devant l'INPI pour les grandes entreprises, et 318 euros pour les plus petites. Les taxes de maintien en vigueur sont de plus de 1 000 euros par an auprès de l'OEB, contre 57 euros à 114 euros devant l'INPI. Enfin, la durée moyenne d'instruction des demandes de brevet devrait, certes, légèrement augmenter, mais les délais de délivrance de brevets devraient être maîtrisés pour toutes les entreprises qui jouent le jeu, c'est-à-dire celles qui déposent un brevet dont l'objectif est de défendre une innovation. En réalité, pourquoi certains s'opposent à ce que les pouvoirs publics renforcent la qualité des brevets français ? Certaines entreprises, souvent les plus grosses, utilisent ce système des brevets faibles et pas chers pour déposer beaucoup de brevets, souvent sans grande valeur, mais qui permettent de bloquer l'arrivée de concurrents. En effet, la PME concernée n'osera pas intenter des recours devant la justice en raison des coûts. Ainsi, faire la promotion d'un brevet faible et pas cher, c'est pénaliser les PME et les start-up en maintenant un rapport de forces qui leur est défavorable. Finalement, elles ne sont pas incitées à innover. Excellente

Une telle disposition législative fragiliserait fortement le système de brevet français, dès lors qu'un risque d'opposition systématique et sans filtre serait théoriquement envisageable. Si le renforcement de la sécurité et de la protection des brevets français est une nécessité pour les PME, ce droit d'opposition engendrerait pour les déposants des coûts administratifs importants, entre les taxes de dépôt, d'enregistrement, d'examen, etc. Un tel dispositif constituerait un frein potentiel à la dynamique de recherche et à la valorisation des innovations françaises, dès lors que les nouveaux coûts induits par cette procédure d'opposition décourageraient les entreprises françaises de protéger leurs innovations sur leur propre marché. Le système de brevet français est aujourd'hui simple et attractif du point de vue financier. Cette modification pourrait conduire certaines entreprises à abuser de ce système d'opposition. Par ailleurs, il faut savoir qu'un droit d'opposition judiciaire existe déjà en France. Le risque de cette nouvelle procédure, je le répète, serait de dissuader les entreprises de déposer des brevets dans notre pays.

Mon cher collègue, je reste un peu perplexe devant l'exposé des motifs de votre amendement, qui me paraît contradictoire. En effet, vous craignez un risque d'opposition systématique tout en redoutant que les coûts induits par cette procédure ne découragent les entreprises de protéger leurs innovations. En ce qui me concerne, je constate qu'il n'existe à l'heure actuelle qu'une seule procédure devant le juge. Elle effraie les PME et les empêche de se défendre, non pas seulement face à leurs concurrentes également PME, mais aussi face à des grands groupes, qui profitent de cette inégalité des entreprises devant la justice selon leur taille.

? En effet, cet article 42 A complète le dispositif en étendant aux dessins et aux modèles ce que l'actuel projet de loi instaure pour les marques et les brevets et auquel nous ne sommes pas, les uns et les autres, opposés. opposés. Mon cher collègue, vous vous inquiétez de la capacité de l'INPI à gérer ces nouvelles missions. Je vous rappelle qu'un délai de deux ans après la promulgation de la loi a été prévu pour l'entrée en vigueur de cette disposition, afin de laisser aux équipes de cet organisme le temps de monter en compétences. Vous évoquez une éventuelle réforme de la directive sur la protection juridique des dessins et modèles de 1998. Or la Commission n'a même pas encore publié

Actuellement, une invention doit obéir à trois critères pour être brevetable : elle doit être nouvelle, elle doit impliquer une activité inventive et elle doit être susceptible d'application industrielle. Or, contrairement à la plupart des offices nationaux de propriété industrielle, l'INPI ne peut pas considérer l'absence d'activité inventive comme un motif de rejet dans le cadre de la brevetabilité d'une invention. Cette spécificité française date des années soixante. À une époque où l'innovation ne constituait pas la clé de voûte de l'économie française, on a privilégié un dispositif qui permettait aux entreprises de disposer assez rapidement d'un titre de propriété pas cher, même s'il ne valait pas grand-chose. ans après, les choses ont évolué et cette exception française est devenue pénalisante pour nos entreprises. Dans une économie dominée par l'immatériel, la compétitivité des entreprises françaises repose de plus en plus sur leur capacité à innover. Mais l'innovation coûte cher et n'est considérée par les entreprises que si elle peut être protégée et valorisée. Cela passe donc par un environnement juridique et institutionnel favorable à la création et à la protection de l'innovation. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas le choix de nombre d'entre vous, mes chers collègues, de défendre la suppression de cet article et, par là même, de maintenir la France dans un système de protection des titres de propriété médiocre, qui nuit à l'essor de nos PME et à leur notoriété. Alors, oui, c'est un véritable changement de mentalité que nous demandons à nos entreprises et à leurs conseils : arrêtons la solution de facilité d'un brevet faible, qui incite les PME à faire l'économie d'une stratégie sérieuse de brevet et aboutit à la délivrance de titres qui ne sont pas opposables On nous dit que le renforcement de la qualité des brevets sera contreproductif pour les entreprises françaises et on nous vante le système actuel. Soyons sérieux : si le système de brevets français était si performant que cela, nous aurions certainement plus d'entreprises innovantes que nos entreprises renonceront au brevet français au profit du brevet européen parce que les coûts seront identiques. C'est faux ! Le brevet français restera avantageux financièrement- chiffres ont été précédemment donnés. En revanche, le renforcement de sa qualité permettra à l'entreprise qui souhaiterait s'étendre à l'étranger d'accéder plus facilement et à moindre coût au brevet européen dans la mesure où elle aura déjà pu prouver le caractère inventif de son invention devant l'INPI. ce que je constate, c'est que le taux de dépôt de brevets auprès de l'INPI stagne depuis cinq ans. Il apparaît que, dans leurs relations commerciales avec les grandes entreprises, les PME subissent un rapport de force qui leur est défavorable non seulement parce qu'elles ne peuvent pas faire valoir leurs droits en raison de l'insécurité juridique qui pèse sur la valeur de leur titre, mais également parce que le faible coût de dépôt des brevets incite les grandes entreprises à en déposer beaucoup, même s'ils sont contestables, ... Il faut conclure, mon cher madame la présidente ! Pas plus ! Si nous n'adoptions pas le renforcement du brevet, nous verrions déferler vers nous les demandes de brevets chinois

Cette nouvelle procédure visant à introduire un examen d'activité inventive est un alourdissement pour les entreprises tant en matière de coûts, de temps que de complexification et de suradministration. Il me semble nécessaire d'en rester au, c'est-à-dire à la procédure que la France a choisie dans les années : confier à l'Office européen des brevets le système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. D'ailleurs, toutes les entreprises implantées en France seraient touchées, aussi bien les petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, les start-up, sans oublier les grandes entreprises. Si l'INPI doit désormais procéder à un contrôle et systématique du critère de l'activité inventive, cela impose également à l'État d'augmenter les moyens alloués à l'INPI, notamment le recrutement de nouveaux personnels, dans un contexte de déficit public record. Dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des comptes avait d'ailleurs mis en garde le Gouvernement contre l'instauration de cet examen au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activités limité à la France. L'adoption de cette mesure a d'ailleurs été faite au détour d'un amendement sans avoir travaillé à une étude d'impact. J'ajouterai que le comité Innovation et recherche, qui représente officiellement les ingénieurs et scientifiques de France, déplore même qu'aucun représentant des entreprises innovantes ni des inventeurs n'ait été consulté en amont avant de mettre ce thème en examen. Enfin, l'Espagne par exemple, a fait, en 2017, le choix de la mesure qui est portée dans l'article 42. Résultat : la chute des dépôts de brevets a été chiffrée à 30 2018. Le risque est aussi que les entreprises se passent du brevet français pour ne déposer que des brevets européens.

vice-président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, premier technopôle d'Europe -et avons été très directement confrontés à cette question des brevets, qui est une vraie question

mieux articuler la recherche, l'industrie et la commercialisation. Nous avons un retard à rattraper

dans ce sens ? Non, c'est exactement l'inverse ! Pardonnez-moi, mon cher collègue Adnot, sur la porte que nous ouvririons, selon vous, aux Chinois, en l'occurrence, c'est exactement l'inverse que nous ferions

il serait souhaitable de supprimer cet article, de continuer à travailler, puis de faire des propositions pour aboutir à des brevets dont l'attractivité et l'efficacité seraient renforcées.

l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réformer les droits des brevets en créant un examen sur le fond des demandes de brevets à l'INPI. Soyons clairs, une telle réforme mettrait à mal l'équilibre du système actuel, qui est apprécié des innovateurs, particulièrement des PME. Avec cette nouvelle procédure, l'examen sur le fond par l'INPI impliquerait, notamment, le critère d'activité inventive, très difficile à apprécier

on ne simplifie rien ! Cette procédure irait complètement à l'encontre de l'objectif recherché consistant à améliorer l'activité du système français et à le simplifier. Je le répète, elle aurait sans nul doute pour effet de dissuader les innovateurs de déposer leurs demandes de brevets en France. Pour toutes ces raisons, je souhaite la suppression

Par conséquent, l'examen au fond et par l'INPI de la brevetabilité de leurs inventions renforcerait le pouvoir de négociation de ces entreprises et faciliterait la valorisation de leur capital immatériel. immatériel. Le système choisi par la France il y a plus de cinquante ans constitue désormais une exception au niveau européen et, au-delà, à l'échelle mondiale. Nos grands concurrents européens disposent à la fois d'un brevet fort national et de la possibilité d'opter pour un brevet européen sans que leur brevet national ait été délesté par les entreprises.

Ils saturent le marché de propositions de brevets qui ne sont pas forcément valables. Ils empêchent les PME d'être inventives et innovantes et de faire valoir des brevets. Au bout du compte, qui est-ce qui trinque ? C'est l'économie française, c'est la crédibilité de l'innovation française ! Il n'y aurait pas d'étude d'impact ? Mais l'étude d'impact, elle a été faite depuis trente

que l'enjeu est absolument décisif et vital pour les PME. Il est décisif pour la crédibilité des brevets français. Avoir le critère d'inventivité délivré par l'INPI avant, c'est donner de la crédibilité aux brevets français.

et je pense à la réputation française en termes d'innovation. Ce texte étant destiné à l'innovation et à la crédibilité de la recherche française, il est indispensable que ce critère d'inventivité soit délivré par l'INPI. Si certains sénateurs du groupe Les Républicains ne sont pas convaincus, je veux rappeler que le plus fervent avocat de ce dispositif à l'Assemblée nationale, celui qui s'est battu pour que le critère d'inventivité soit reconnu par l'INPI, c'est le député Les Républicains Daniel Fasquelle, qui a indiqué que c'était probablement l'une des meilleures propositions du texte.

Il faut penser aux conséquences qu'aura l'instauration de l'analyse de l'activité inventive. Cette activité est somme toute assez mystérieuse : on ne sait pas très bien ce que c'est.

probablement une centaine d'examinateurs. Enfin, je rappelle que le choix français a été l'intégration dans le système européen. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

Éric Carreel, dirigeant de Withings, Sculpteo, Invoxia et Zoov. Bref, nous avons fait notre travail de parlementaire, qui consiste, d'une

Sinon, tout ce travail législatif serait inutile. Je pense pour ma part avoir montré, depuis le début de l'examen de ce texte, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que j'étais ouvert à toutes les propositions d'amélioration.

monsieur Daunis, sur des propos que j'aurais tenus à ce micro. Je maintiens ce que j'ai dit, monsieur le sénateur, et je pense pour le coup que ce n'est pas de bonne politique que d'aller expliquer que le ministre raconte des choses fausses

le sénateur, sont têtus ! Il se trouve que la France a le taux d'annulation de ses brevets le plus élevé de tous les pays européens. Cela devrait tous nous interroger ! Il ne s'agit pas de savoir qui va l'emporter et qui va perdre dans cette affaire

ont choisi d'assurer l'examen de l'inventivité des brevets afin de garantir la solidité de l'innovation. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des autres pays européens, et c'est le cas des grands pays asiatiques, au premier rang desquels la Chine. Je veux bien qu'on persiste à défendre un dispositif dans lequel nous sommes les seuls à nous y retrouver, mais j'estime qu'il n'est pas mauvais de regarder ce que font nos voisins et d'essayer de trouver une solution qui soit plus efficace afin de légitimer, de consolider et de valoriser l'innovation française. Enfin, je salue la sagesse du sénateur Alain Richard et je suis très favorable à sa proposition. S'il y a encore débat sur le sujet, je propose que nous nous mettions autour d'une table, que nous échangions nos arguments sur le sujet, que nous examinions les difficultés qui peuvent encore se poser et que nous essayions de trouver un compromis sur la reconnaissance préalable du critère d'inventivité des brevets français pour améliorer la qualité de l'innovation française. Cela suppose simplement- techniquement, à mon sens -que les amendements déposés soient retirés et que nous nous retrouvions pour en discuter. J'y suis évidemment extrêmement favorable.

dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leur patrimoine immatériel protégeable : brevets d'invention, marques, droits d'auteur, dessins et modèles. Certaines des missions des conseils en propriété industrielle sont exercées conjointement avec des avocats. Il existe pourtant des différences de réglementation entre les deux professions, alors même que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s'associer au sein des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice

l'obligation suivante : les conseils en propriété industrielle ou assimilés devront détenir, ensemble, au moins la moitié du capital et des droits de vote des cabinets de conseil en propriété industrielle. Il s'agit d'éviter toute interférence due à la présence d'un fonds de pension, ou de toute autre structure financière, et de défendre ainsi au mieux les intérêts des innovateurs et, plus particulièrement, des PME.

Or il existe des différences de réglementation entre les deux professions. Ainsi, en l'état actuel, les garanties de confidentialité des conseils en propriété industrielle sont inférieures à celles qui

d'une part, en autorisant l'officialisation des courriers entre conseils en propriété industrielle, ou entre un tel conseil et un avocat ; d'autre part, en précisant que la confidentialité d'une correspondance entre un conseil en propriété industrielle et un avocat doit être respectée de manière identique,

Jean-Marc Gabouty. Cet amendement tend à harmoniser et à clarifier les règles de prescription des actions en contrefaçon et d'atteinte au secret des affaires, ainsi qu'à rendre imprescriptible l'action en nullité des titres de propriété industrielle. S'agissant des actions en contrefaçon, le point de départ du délai de prescription serait non plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon, mais celui où le requérant a eu connaissance, ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance, du dernier fait justifiant l'action, conformément à l'esprit du code civil et des textes européens. Cette disposition allonge le délai pour agir en contrefaçon, en permettant d'engager une action tant que la contrefaçon se poursuit et de viser des faits ayant débuté plus de cinq ans auparavant, alors que cette réparation est aujourd'hui Cela permettrait de renforcer la lutte contre la contrefaçon et d'améliorer l'indemnisation des préjudices résultant des faits de contrefaçon. La même modification est apportée dans le code de commerce en ce qui concerne la prescription de l'action relative à une atteinte au secret des affaires, dans un souci de cohérence. S'agissant des actions en nullité, au vu du silence du code de la propriété intellectuelle sur ce point, les juridictions appliquent la prescription de droit commun, à savoir cinq ans depuis la réforme de 2008. Cette solution conduit à empêcher, au-delà d'une courte durée, la remise en cause d'un titre affecté d'un vice intrinsèque, bloquant abusivement un marché pour de nouveaux entrants, ou portant atteinte à l'ordre public. En outre, la situation actuelle est source d'une grande insécurité juridique, les juridictions ayant des appréciations divergentes du point de départ du délai de prescription de cinq ans. L'absence de prescription de l'action en nullité permettra d'assainir la concurrence, en éliminant les titres nuls, et de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public.

du XXI siècle. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, même si je regrette qu'une réforme aussi fondamentale soit engagée à l'occasion d'un simple amendement en séance publique.

Le développement des nouveaux usages de la route conduit à prévoir la restriction à certaines catégories de véhicules de l'accès à tout ou partie de la voirie. De telles pratiques se sont développées depuis de nombreuses années

L'amendement que je vous propose d'adopter vise, d'une part, à développer de nouveaux usages favorisant la performance des transports en commun et la lutte contre la congestion routière de manière à réduire la pollution et, d'autre part, à faciliter les expérimentations de véhicules autonomes sur des itinéraires dont l'aménagement aura été préalablement réalisé par la puissance publique.

de mieux gérer le trafic routier. Toutefois, cela me paraît un peu prématuré. Par ailleurs, le nombre de véhicules autonomes ne justifie pas aujourd'hui qu'on bloque une voie d'autoroute

d'autoconsommation ont vu le jour. Nous sommes là, évidemment, bien loin des objectifs que nous nous sommes fixés. Heureusement, nous ne légiférons pas pour 6 projets sur tout le territoire national ! De nombreux acteurs appellent donc à une simplification.

municipal équipé ne pourrait pas alimenter un autre bâtiment municipal du fait de ce critère fondé sur le poste de transformation électrique. Voilà la situation à laquelle cet amendement vise à répondre.

dessus dès à présent paraît donc pour le moins prématuré, au vu du faible recul que nous avons sur des pratiques qui sont encore embryonnaires.

Il faut aussi savoir que l'autoconsommation collective permet de déroger à certaines règles de protection des consommateurs. C'est d'ailleurs pourquoi la Commission de régulation de l'énergie elle-même a recommandé, en février 2018, de s'en tenir au périmètre actuel. Il y a donc clairement un risque de remise en cause des principes de solidarité et d'équité entre les usagers et les territoires. On risque aujourd'hui d'aboutir, peut-être rapidement, à une forme d'individualisme ou de communautarisme énergétiques. D'où la nécessité d'encadrer ces pratiques et de ne pas dessaisir le législateur de ces sujets. Absolument ! C'est la raison pour laquelle je confirme ici l'avis défavorable de la commission

Par exemple, la personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation n'est pas soumise à l'obligation d'informations précontractuelles en matière de contrat de fourniture de l'électricité, à celle de proposer un contrat d'une durée d'un an ou de respecter les dispositions relatives à la facture. Elle n'est pas non plus soumise à l'obligation de vendre l'électricité à un prix identique à tous, ce qui déroge au principe de péréquation tarifaire. Le consommateur dispose-t-il du droit de résilier un contrat sans frais, à tout moment ? C'est une autre question. Pourra-t-il utiliser le chèque énergie pour payer le producteur local ? Bref, faut-il dès à présent aller dans le sens de l'amendement du Gouvernement alors qu'il existe peu peu de retours d'expérience sur le fonctionnement réel de ces opérations ? Je rappelle qu'en janvier 2019 seules 10 opérations étaient en service, regroupant un total de 47 consommateurs. Dès lors, monsieur le ministre, pourquoi ne pas mettre en place des expérimentations ciblées- je dis bien ciblées -d'élargissement du périmètre ? Cela permettrait de disposer d'un retour d'expérience fiable, fiable, à partir duquel nous pourrions décider des obligations qui doivent, à terme, s'appliquer aux opérations d'autoconsommation collectives et du périmètre pertinent au vu de ces obligations. Je suis favorable à l'autoconsommation et à son développement, mais toutes ces interrogations me troublent. N'est-ce pas prématuré d'aller très vite ... trop vite ? Très bien ! La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

La séance est reprise. Mes chers collègues, je viens d'adresser à Mme le maire de Paris et à Mme le maire du XVI arrondissement les pensées du Sénat

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site

Territoires. Madame la ministre, comme vous le savez, les États-Unis ont décidé vendredi dernier de suspendre leur participation au traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, Ils justifient leur position du fait que les Russes seraient sur le point de mettre en place de nouveaux missiles, en violation du traité. Ce traité concerne particulièrement l'Europe, puisqu'il trouve son origine dans la crise des euromissiles des années 1970. À cette époque,

bilatéral signé par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev permette de supprimer cette catégorie de missiles des deux côtés. Autre inquiétude Vladimir Poutine a indiqué un vice-ministre que le traité de réduction des arsenaux nucléaires, qui arrive à terme en 2021, pourrait ne pas être reconduit.

L'Europe doit pourtant prendre ses responsabilités à l'égard d'un allié qui ne se montre pas toujours fiable et prévisible, et à l'égard d'une Russie qui multiplie les coups de force pour affirmer sa puissance. quelle initiative comptent prendre la France et ses alliés européens pour éviter le risque d'une nouvelle course aux armements nucléaires ? La parole est

Des armes nucléaires américaines et soviétiques stationnées sur le sol européen, par leur portée, ne pouvaient frapper que l'Europe. C'est à ce péril qu'est venue mettre fin la signature, en 1987, du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui engageait l'élimination de ces armes de notre continent. Aujourd'hui, ce traité est remis en cause par les Russes qui en violent les règles et par les Américains qui annoncent vouloir s'en retirer. La Russie a immédiatement fait savoir qu'elle voulait développer un nouveau missile. Nous sommes dans une situation paradoxale. Les Européens ne font pas partie du traité FNI, mais c'est bien de la sécurité de notre continent qu'il s'agit. Nous sommes devant un risque de relance de la course aux armements, mais aussi devant un nouvel épisode d'attaque en règle contre le multilatéralisme. Alors, que faut-il faire ? Tout d'abord, et nous le faisons, il faut appeler la Russie à répondre aux demandes qui lui ont été adressées et à remplir pleinement ses engagements. Dans le même temps, et vous le rappelez, il convient de construire une véritable autonomie stratégique européenne. L'Europe de la défense a plus progressé en deux ans qu'en six décennies. Le fonds européen de la défense est désormais en place. La coopération structurée permanente est lancée ; elle rassemble vingt-cinq États. Nous avons également besoin de l'initiative européenne d'intervention, que nous avons engagée et qui permet de créer une culture stratégique commune entre les Européens les plus capables et les plus volontaires. Prenons garde de croire que les traités de maîtrise des armements appartiendraient à l'histoire et seraient dépassés. Dans le contexte international incertain que nous connaissons, ils sont plus indispensables que jamais. Nous appelons ainsi la Russie et les États-Unis à prolonger au-delà de 2021 le traité New START sur les arsenaux nucléaires et à négocier le traité successeur. Si nous voulons éviter de voir régner la loi du plus fort au péril de notre sécurité, nous devons continuer à veiller à la force de la loi. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour le groupe Les Républicains. Républicains. Monsieur le Premier ministre, un référendum le jour des élections européennes Les pauvres, elles n'avaient rien demandé ! Pour répondre à des manifestants d'hier et d'aujourd'hui qui dénoncent trop d'impôts, trop de taxes, pas assez de pouvoir d'achat, une dépense publique à revoir, trop de contraintes réglementaires,

La question que vous posez me semble parfaitement légitime puisque la Constitution, vous le savez, prévoit en son article 11 la possibilité que le Président de la République soumette au référendum un certain nombre de projets de loi. Cette procédure a été utilisée huit fois depuis 1958 pour trancher des questions importantes sur l'avenir du pays.

Au moment où nous parlons, monsieur le sénateur, plus de 4 000 réunions ont déjà eu lieu, plus de 700 000 contributions ont été déposées sur le site. Je ne comprends pas pourquoi vous sifflez, ce sont des chiffres réels, c'est tout Je crois donc, monsieur le sénateur, qu'il convient de laisser ces débats se dérouler. Vous le savez, le Président de la République et le Gouvernement sont à l'écoute des Français. Mais oui Mais oui ! J'ai moi-même eu l'occasion de me rendre dans une petite commune du Tarn, à Giroussens, où les gens se respectaient et évoquaient, dans le calme et la fermeté, ce qui traçait, pour eux, les lignes directrices de leur avenir. Une fois ce grand débat achevé, il faudra en tirer les conséquences, cela a été clairement dit, de manière précise et concrète. Il appartiendra alors au chef de l'État et au chef du Gouvernement de faire les choix qui s'imposeront.

pour la réplique. Je vous rassure, madame la ministre, je n'ai aucune appréhension par rapport à un référendum. Je pense que le Président de la République en aurait davantage.

! Je veux bien tous les grands débats, mais j'ai entendu le Président de la République dire que, ce qui compte, c'est tout de même ceux qui ont été élus. Monsieur le Premier ministre, 348 sénateurs, 577 députés, 925 parlementaires, 925 citoyens : rien. Mais 348 sénateurs, 577 députés, 925 parlementaires élus de manière directe ou indirecte : c'est la France ! La parole est à M.

ce qui apparaît dans les conclusions de ce débat pour présenter des réponses sous une forme ou sous une autre. Notre collègue Roger Karoutchi vient de le rappeler, le Parlement le Parlement est fait pour cela et il est disponible pour discuter des réponses susceptibles d'être apportées à tous ceux qui débattent aujourd'hui. Le Parlement ne s'use que si l'on ne s'en sert pas Il est donc indispensable, effectivement, de présenter devant l'Assemblée nationale et le Sénat les propositions qui pourront être portées par la voie législative. Le chef de l'État et le chef du Gouvernement peuvent aussi utiliser une autre voie, Mme le garde des sceaux vient de le rappeler : elle est prévue par la Constitution, elle est légitime, c'est celle du référendum. Si tel était le cas,

Il est indispensable que nous puissions avoir un vrai débat sur la construction européenne. L'Europe est en crise, l'Europe est malade. Nous voyons jour après jour les soubresauts attristants du Brexit.

retrouve le rôle moteur qui doit être le sien en Europe et que nous puissions avoir ce débat. Évitons, pour cela, d'organiser un référendum le jour des élections européennes

On peut toujours, ici ou là, dire que telle ou telle réunion ne ressemble pas à ce que l'on aurait souhaité dans l'idéal. Toutefois, les réunions sont nombreuses, elles interviennent dans de grandes villes comme dans de toutes petites communes et elles permettent à nos concitoyens de s'exprimer.

j'en suis intimement convaincu. Tout ce qui aurait pour effet de remettre en cause la clarté du débat serait probablement à écarter. C'est d'autant plus vrai que, référendum ou pas, monsieur le sénateur, depuis très longtemps, lors des élections européennes,

Je rappelle aussi que la France est l'un des derniers pays au monde à mettre en place le prélèvement à la source, qui existe depuis 1920 dans beaucoup de pays, et depuis 1945 partout en Europe. Seule la Suisse ne l'a pas adopté. Sauf pour

Il n'y a aucun bug technique ou systémique et la décision prise par le Premier ministre en juillet 2017 de reporter l'application d'un an nous a permis, à Gérald Darmanin et moi-même, de régler un certain nombre de questions, notamment pour les particuliers employeurs ou sur le versement d'un acompte de 60 % pour les crédits d'impôt. Cette réforme, nous l'accomplissons d'abord pour les Français, car elle nous permettra d'adapter l'impôt aux revenus de nos concitoyens, avec une véritable contemporanéité du prélèvement. C'est d'autant plus important que 7 millions de nos concitoyens connaissent chaque année une variation de leurs revenus d'au moins 30 %. Nous pourrons ainsi faire en sorte qu'ils soient assujettis de la manière la plus juste qui soit. Nous engageons aussi cette

Le premier jour, 500 000 contribuables ont, d'une manière ou d'une autre, contacté les services fiscaux. Depuis le début du mois de janvier, nous avons modifié le taux de plusieurs centaines de milliers de contribuables pour mieux tenir compte de la réalité de leurs revenus. Nous avons fait en sorte que cette réforme fonctionne bien et qu'elle fonctionne aussi avec les collecteurs, à savoir les entreprises, qui peuvent constater aujourd'hui que la mise en oeuvre se fait dans de bonnes conditions et à un coût bien moindre que ce qu'elles pouvaient craindre.

Alors que la consommation de tabac baisse globalement dans notre pays, certains territoires demeurent malheureusement en marge de cette dynamique positive. Si les causes sont assurément multifactorielles- on fume davantage en situation socio-économique défavorable -, l'une des explications est aussi géographique. En effet, les quatre régions où l'on trouve le plus de fumeurs- PACA, Hauts-de-France, Occitanie et Grand Est -sont proches de pays où le tabac est le moins cher. Avec un paquet de référence à 5,40 euros, le Luxembourg attire les fumeurs du Grand Est en quête de cigarettes à moindre coût, notamment ceux du Nord lorrain où les taux d'incidence du cancer du poumon sont significativement plus élevés que la moyenne nationale. D'après une récente étude de Santé publique France, les départements frontaliers de la région présentent les situations les plus préoccupantes. Et pour cause : l'augmentation du prix du tabac en France, mesure que j'ai soutenue et qui a fait la preuve de son efficacité, a malheureusement encore renforcé ce différentiel entre les zones transfrontalières et le reste du territoire. Face à ce constat, la région Grand Est a lancé un programme de lutte contre le tabac. le tabac. Cibler les publics les plus à risque doit en effet être au coeur de toutes les politiques de prévention et d'accompagnement. Néanmoins, la forte attractivité de nos voisins doit absolument être prise en considération par le Gouvernement pour chaque action entreprise, sous peine de voir se renforcer les inégalités territoriales en matière de santé.

vous avez eu raison de poser d'emblée votre question à Agnès Buzyn, car c'est aussi une manière de souligner l'implication de Mme la ministre de la santé dans la lutte contre le tabac et ses conséquences sur la santé publique. Toutefois, le fond de votre question concerne essentiellement l'impact du trafic de tabac, et parfois même de la contrebande, en matière d'action publique. Vous nous interrogez sur les actions que mène le Gouvernement pour diminuer les trafics de tabac dans les zones frontalières. Nous avons pris un certain nombre de dispositions, notamment à l'occasion de l'adoption de la loi de lutte contre la fraude, la fraude, en abaissant de 10 à 4 le nombre de cartouches qui peuvent être importées d'un pays de l'Union européenne pour faire en sorte que, au-delà de 4, il y ait une présomption de contrebande permettant à nos douaniers de pouvoir sanctionner celles et ceux qui se livrent à ces trafics de proximité. Nous avons aussi fait en sorte de doubler les amendes pour trafic frontalier en matière de trafic de tabac, en passant l'amende maximale de 2 500 euros à 5 000 euros afin de dissuader les trafics que vous pointez. Au-delà, nos services sont mobilisés de manière massive. Depuis trois ans, 1 500 tonnes de tabac ont été saisies. Pour prendre un exemple que vous connaissez bien, le 27 septembre dernier, à Saint-Avold, c'est 1,2 tonne de tabac qui a été saisie à l'occasion d'un contrôle inopiné. Nous développons de nouvelles techniques de ciblage pour faire en sorte d'agir avant le dédouanement et nous contrôlons aussi de plus en plus souvent des lieux de vente ou de trafic situés au-delà des frontières, mais dont on sait qu'ils sont propices à cette consommation de tabac. Enfin, nous avons ouvert des discussions avec nos partenaires européens. Nous souhaitons tout d'abord revoir la directive de 2011, qui fixe des minima fiscaux en matière de tabac, de manière à aller vers l'harmonisation fiscale que vous appelez de vos voeux.

plus précisément sur les conditions d'exercice du pluralisme dans ce débat politique et médiatique. Déjà, vous voulez restreindre la liberté de manifester.

aux Français ou à une campagne présidentielle de rattrapage dans laquelle il n'y aurait cette fois qu'un seul candidat ? En matière de temps de parole, les compteurs du CSA doivent exploser. Il serait d'ailleurs intéressant que les chiffres soient publiés au fil du débat, et pas dans trois mois Et rien ne s'arrangera avec les élections européennes, puisque la loi que vous avez fait voter va répartir les temps de parole de manière scandaleusement inégale. inégale. Ma question est la suivante : quelles mesures comptent prendre le Gouvernement et les garants pour assurer, jusqu'au terme de ce débat et ensuite, une égalité d'accès au temps de parole politique et médiatique, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui ?

qui ont été nommés par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président du Conseil économique, social et environnemental et par le Gouvernement. Ces cinq personnes nous aident à respecter les principes que nous nous sommes fixés.

Son encre est à peine sèche. Pourtant, les ordonnances qu'elle vous a autorisés à rédiger suscitent de vives inquiétudes dans le milieu agricole, notamment chez les trois quarts des agriculteurs membres d'une coopérative, qui craignent une remise en cause du statut coopératif. En effet, vos ordonnances assimileraient les coopératives à des entreprises commerciales pour le calcul du prix d'achat aux agriculteurs. Ce prix- c'est tout l'objet de la loi Égalim -ne doit pas être abusivement bas au regard d'indicateurs à préciser. Monsieur le ministre, il faut comparer ce qui est comparable. La coopérative est la continuité de l'exploitation, et non une entreprise commerciale. L'inquiétude dont je me fais le porte-voix vient de ce que la notion de prix serait appliquée par votre ordonnance aux relations entre la coopérative et l'adhérent. Or la coopérative, jusqu'à présent, n'achète pas le produit, mais le vend aux entreprises commerciales. C'est aussi pour cela que le médiateur de la coopération agricole ne doit pas être remplacé par un médiateur de la relation commerciale. Certes, il peut y avoir des abus dans certaines grosses coopératives, dont la gouvernance est assez éloignée des adhérents. Il faut évidemment les corriger, mais pas au prix d'une remise en cause de la singularité du modèle coopératif, qui est fondé sur l'humain et la solidarité. Beaucoup d'exploitations sont de taille modeste, notamment en Occitanie, comme me le souffle mon collègue du Gers, Franck Montaugé, que j'ai plaisir à associer à cette question. Elles sont fragiles, mais elles font vivre les territoires, le modèle coopératif étant un outil performant pour une agriculture saine et de qualité. Certains pensent qu'à terme l'objectif de Bercy serait de parvenir à fiscaliser le chiffre d'affaires des coopératives, ce qui reviendrait à taxer deux fois les coopérateurs. Monsieur le ministre, nous connaissons votre attachement à l'agriculture et aux agriculteurs. les défendre non pas seulement contre les critiques, mais aussi contre les logiques purement économiques, qui leur sont défavorables. Ma question est simple : quelles preuves de soutien vos ordonnances apporteront-elles à notre modèle coopératif agricole ? La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Les services du ministère de l'agriculture travaillent en étroit partenariat avec les représentants des coopératives, y compris sur la rédaction de cette ordonnance. Et avec le Parlement ? Le prix abusivement bas est effectivement par nature et par construction une notion juridique qui peut entrer en contradiction avec la construction d'un prix coopératif. C'est pourquoi l'ordonnance veille à préserver le modèle coopératif en maintenant, dans le code rural et non dans le code de commerce- ce n'est pas un point négligeable -la notion de prix abusivement bas et en instituant le recours au Haut Conseil de la coopération agricole ou au médiateur de la coopération agricole en cas de pré-litige, et non au médiateur des relations commerciales. Nous voulons maintenir l'excellence de l'agriculture française et le modèle coopératif,

de réduire les niches fiscales en diminuant le plafond global de ces dernières ou en imposant des conditions de ressources pour en bénéficier, afin, dites-vous, monsieur le ministre, qu'elles profitent aux classes moyennes plutôt qu'aux classes La fiscalité française est un objet de curiosité qui place la France au premier rang des pays européens dont l'impôt est le plus lourd. Les deux ans que vous avez passés à Bercy n'y auront rien changé. Ce sont ces fameuses niches fiscales qui offrent une bouffée d'oxygène aux contribuables écrasés par l'impôt. Aujourd'hui, la crise des « gilets jaunes » et le besoin de ressources supplémentaires conduit votre gouvernement à raboter ces niches, l'objectif étant de montrer du doigt ces contribuables qui bénéficient de niches fiscales pour les désigner comme des privilégiés. Soudain, ces mécanismes dont on vantait l'utilité- emplois à domicile, dons aux associations, investissements dans la transition énergétique -n'auraient plus aucune justification. Monsieur le ministre, clairement, vous gérez une crise politique née d'un ras-le-bol fiscal en créant tout bonnement une nouvelle hausse d'impôt ! Eh oui ! Voilà encore une mesure à l'encontre des classes moyennes Quand allez-vous cesser de matraquer ces Français qui travaillent, payent des impôts et assurent la solidarité nationale ? comptes publics. Madame la sénatrice, vous nous interrogez sur la dépense fiscale et je me dois avant tout d'excuser Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, qui est retenu par Vous annoncez, dans votre question, que nous aurions décidé de revenir sur certaines niches fiscales. Or il n'en est rien, aucune décision n'ayant été prise. En revanche, il est important et intéressant d'ouvrir ce débat. La dépense fiscale peut être un bon levier pour promouvoir des comportements vertueux ou inciter à tel ou tel investissement en direction de l'emploi ou de diverses politiques publiques.

Nous allons travailler sur ce sujet avec en tête deux impératifs. Le premier est de continuer ce que nous faisons depuis le début, c'est-à-dire diminuer les prélèvements obligatoires sur les ménages et, en aucun cas, taxer les classes moyennes. Allons ! Le deuxième vise à renforcer l'égalité. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu,

Le déficit public, qui devait être contenu sous la barre des 3 %, est annoncé à 3,3 % en 2019. Quant au taux de prélèvements obligatoires, que vous estimiez à 44,3 % dans la loi de programmation, il atteindra 45 % du PIB. Il n'y a pas de quoi pavoiser, monsieur le secrétaire

de la recherche et de l'innovation. Madame la ministre, dans un monde en pleine transformation technologique, l'investissement dans la recherche constitue plus que jamais un enjeu capital pour notre pays. Malgré une légère amélioration, la France, qui, avec les autres pays de l'Union européenne, s'était fixé pour 2020 un objectif de recherche globale de 3 % de son PIB,

et même si aucun chiffre précis n'a encore été avancé, l'annonce par M. le Premier ministre, voilà quatre jours, d'une future loi de programmation pluriannuelle pour la recherche est déjà, en soi, une excellente nouvelle.

par la France, et aux côtés de l'Union européenne, ne peut qu'être favorable au renouveau de nos industries, à la compétitivité de notre économie, ainsi qu'à notre souveraineté numérique. Madame la ministre, pourriez-vous aujourd'hui nous préciser quelles seront les priorités de cette programmation et comment elles seront articulées avec les mesures du prochain cadre pluriannuel financier européen, couvrant les années 2021 à 2027 ? Enfin, dans la phase de concertation et de préparation de la future loi qui va s'ouvrir, comment entendez-vous mobiliser au mieux la communauté scientifique, les industriels et l'ensemble de la communauté nationale sur ce sujet ? La parole

bien longtemps, trop longtemps même, qu'un chef de gouvernement n'avait pas souhaité réaffirmer, devant la communauté scientifique, combien nous lui faisons confiance pour améliorer l'avenir de notre pays,

souvent, nous ont empêchés d'avancer sur les questions de recherche, notamment les oppositions stériles entre la recherche publique et la recherche privée- partout dans le monde, on parle de recherche -et la compétition stérile entre les financements compétitifs et les financements récurrents-

les activités de recherche de base, celles des laboratoires, et une recherche compétitive de qualité, sans risque d'exclure certains excellents projets

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre, s'il veut bien me répondre. Monsieur le Premier ministre, les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont voté hier la même délibération, demandant la création d'une nouvelle collectivité territoriale : la « collectivité européenne d'Alsace C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, celui de l'entrée dans un processus législatif qui pourrait conduire, je l'espère, à la renaissance de la région Alsace. Ce sont aussi des nouvelles questions qui se posent : quelles compétences seront en définitive dévolues à cette collectivité ? En effet, dans l'état actuel de nos connaissances, le projet de loi qui doit en préciser les termes reste largement insatisfaisant. Non seulement il ne décline pas entièrement les compétences figurant dans la déclaration de Matignon du mois d'octobre dernier, mais il ne dit rien de celles qui pourraient être transférées de la région Grand Est. Je voudrais rappeler, ici, que 84 %, puis 83 % des Alsaciens ont indiqué, dans deux sondages successifs, vouloir retrouver une collectivité régionale alsacienne de plein exercice. Pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, nous éclairer ? Cependant, mes chers collègues, le choix des Alsaciens illustre une question plus générale, que les maires ont posée de façon récurrente au Président de la République. Ces derniers en ont assez de la recentralisation rampante ; ils en ont assez des contraintes ; ils veulent plus de liberté, de souplesse ils souhaitent que les périmètres des collectivités ne soient plus déconnectés des réalités économiques, sociales et culturelles des territoires. La loi du 7 août 2015 portant

La démocratie participative peut parfois être une réponse, mais, dans ce domaine de la réforme territoriale, on doit pouvoir faire confiance à la démocratie représentative.

du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour la constitution d'une nouvelle collectivité territoriale. Vous l'élargissez, ensuite, pour évoquer les limites du dispositif issu de la loi NOTRe et les correctifs qui pourraient y être apportés.

de décisions ayant d'ailleurs été prises bien avant la nomination de ce gouvernement. Ayant entendu ces interrogations, ayant d'emblée fixé une limite, formulée par le Président de la République durant la campagne présidentielle, de non-remise en cause des périmètres régionaux tels qu'ils avaient été décidés, nous avons essayé

que nous sommes parvenus à une déclaration commune avec le président du conseil régional, avec les deux présidents des conseils départementaux, avec de très nombreux parlementaires. Cette déclaration commune, signée à Matignon,

Celui-ci aura l'occasion de se prononcer sur un très bel exemple de coopération intelligente entre les élus locaux, les parlementaires et le Gouvernement. Je ne prétends pas que tout est réglé par cette déclaration commune. peut-être est-ce votre cas ? -, vous l'avez dit vous-même, monsieur le sénateur, veulent aller plus loin, d'autres veulent aller beaucoup moins loin. Mais je pense que nous avons progressé, et ce en écoutant et en inscrivant dans le dispositif juridique quelque chose qui peut faire consensus. Partant de cette méthode, qui n'est pas propre à l'Alsace, car nous l'avons reproduite dans d'autres territoires, vous estimez qu'il convient de modifier ce que l'on appelle parfois les « inconvénients » de la loi NOTRe, parfois ses « irritants ». Il en

au détriment de ce qui aurait pu se construire dans de bonnes conditions dans certains territoires. C'est un équilibre délicat, qui exigera beaucoup de finesse et de travail. Je suis certain que le Sénat et le Gouvernement travailleront dans d'excellentes conditions, ensemble, sur le sujet.

ministre, vous en attaquez les fondements constitutionnels : le bicamérisme tout d'abord- nous sommes au Sénat -, que le Président de la République a mis en cause ouvertement dans sa lettre aux Français, mais aussi la liberté d'aller et venir, et le droit de manifester désormais sous une chape préfectorale par votre loi « anticasseurs Vous vous attaquez également, depuis des mois, à la liberté de l'information, avec la loi sur le secret des affaires, puis la loi sur les fragilisant le travail des journalistes, la protection des sources et les lanceurs d'alerte. Le Président de la République voudrait aujourd'hui créer des structures subventionnées devant veiller à la neutralité de l'information, au parfum de Pravda ou d'ORTF ! Ces mesures, ces déclarations font système ensemble et doivent nous alerter. Hier, c'était une tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart à laquelle nous avons assisté, inédite et inquiétante parce qu'elle touche à la protection des sources. Cet événement éclaire d'un jour édifiant votre attention particulière à la nomination de procureur de Paris et votre refus de l'indépendance du parquet. Monsieur le Premier ministre, votre majorité joue un jeu dangereux ! On ne joue pas avec les libertés publiques ! Le paysage démocratique qui se dessine sous nos yeux inquiète, y compris dans les rangs de cette majorité- il suffit de voir le score du vote sur la loi anticasseurs. Quand allez-vous cesser de fragiliser nos libertés fondamentales ?

portant sur des infractions d'atteinte à la vie privée. Deux magistrats de ce parquet se sont donc rendus au journal Mediapart pour se faire remettre les enregistrements sonores de conversations qui seraient intervenues entre MM. Benalla et Crase. Les magistrats agissaient, je tiens à le préciser ici, dans le cadre non coercitif de l'enquête préliminaire, et ne pouvaient pas procéder à une saisie sans l'assentiment du représentant légal de l'entreprise de presse. Mediapart a, dans un premier temps, refusé de remettre ces enregistrements, puis les a donnés à la justice, ce qui permettra de faire toute la lumière sur cette affaire.

Le protoxyde d'azote est devenu le troisième produit psychoactif le plus consommé chez les étudiants français, selon une récente étude de la mutuelle SMEREP. Dans nombre de villes SMEREP. Dans nombre de villes du Nord, par exemple, le sol des espaces publics est aujourd'hui jonché de ces capsules grises de ballons éclatés, qui laissent à penser à une véritable banalisation de l'usage de ce produit par le détournement de son usage conventionnel, que ce soit par le biais de cartouches de gaz pour siphon à chantilly ou de bonbonnes médicales dédiées aux anesthésies. Nouvelle drogue tendance et récréative, le protoxyde d'azote, gaz hilarant, fait donc fureur chez les jeunes, avec une véritable dépendance à l'effet euphorisant, et ce d'autant qu'il est en vente libre, à un coût très modique et sans restriction. Aucun visuel ou pictogramme sur l'emballage n'alerte sur les dangers d'inhalation de ce produit. Bénéficiant d'une réputation de gaz récréatif non addictif, de drogue bon marché ayant une nocivité négligeable, ce produit a donc tout pour plaire ! Pourtant, ses dangers sont bien réels. Le protoxyde d'azote n'étant pas métabolisé par l'organisme, ses utilisateurs se sentent souvent parfaitement normaux dans les deux minutes suivant l'inhalation, ce qui les conduit à poursuivre leur consommation. Mais vertiges, maux de tête, vision floue, malaises, crise de panique, problèmes cardiaques peuvent survenir. La consommation excessive de ce produit a des effets graves sur la santé. Elle a déjà fait de nombreuses victimes en Grande-Bretagne puisque, entre 2006 et 2012, 17 personnes en sont décédées, et 2 cas sont déjà connus en France.

Pour son usage commercial d'aérosol, la réglementation est celle des produits de consommation courante. Compte tenu de l'usage détourné de ces produits de consommation courante, il nous apparaît vain

de la prévention, et ce dès le plus jeune âge, et vous savez à quel point la prévention est au coeur de la politique de ce ministère. Soyez convaincue que nous sommes pleinement engagés pour lutter à vos côtés, aux côtés de tous les élus locaux contre ce phénomène. Nous devons mettre en oeuvre les actions les plus pertinentes, et ces actions passent sûrement, en priorité, par l'école, par les universités, par les acteurs en proximité des jeunes et aussi, peut-être, par les étudiants du service sanitaire- ils sont 47 000 depuis cette rentrée à agir auprès de nos jeunes.

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de

M. le ministre. Cet amendement vise à limiter le champ d'application de l'expérimentation qui est prévue à l'article 43 en excluant le champ spécifique des ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et la maîtrise des risques graves pour la santé humaine.

avant que ne commence le débat sur la privatisation d'Aéroports de Paris, je souhaite vous rappeler quelques données sur cette société qui constitue un actif stratégique unique pour le développement économique et touristique de la Nation et pour sa connectivité avec le reste du monde. Créé en 1945 sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, transformé en société anonyme en 2005, Aéroports de Paris a pour mission d'aménager, d'exploiter et de développer les plateformes franciliennes. En 2017, les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ont pour la première fois franchi, à eux deux, la barre des 100 millions de passagers accueillis, avec un total de 101,5 millions de passagers. L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est à lui seul le dixième aéroport mondial en termes de trafic passagers et le deuxième aéroport d'Europe.

Les aéroports franciliens constituent la principale frontière de la France, elle-même première destination touristique mondiale, avec plus de 90 millions de visiteurs en 2018, et la voie d'accès privilégiée depuis l'étranger à Paris et à la région d'Île-de-France, première région économique française. En conséquence, la capacité d'Aéroports de Paris à fournir un service public de très haut niveau aux compagnies aériennes du monde entier ainsi qu'à leurs passagers est cruciale pour renforcer l'attractivité de notre pays. Elle est également très importante pour l'avenir du pavillon français dans la mesure où la compagnie Air France-KLM représente à elle seule, avec ses partenaires, 50 % de l'activité de Paris-Orly et 62 % de celle de Paris-Charles-de-Gaulle, qui constitue son- chiffres de 2017. Les aéroports parisiens ont naturellement un fort impact sur l'économie de la région d'Île-de-France. On estime ainsi que plus de 122 000 personnes travaillent sur les plateformes aéroportuaires franciliennes. Le nombre total d'emplois engendrés par le système aéroportuaire francilien est estimé à plus de 570 000, soit près de 8 % de l'emploi salarié francilien. Le potentiel de développement de Paris-Charles-de-Gaulle est très important puisque ses quatre pistes pourraient lui permettre d'accueillir à terme entre 140 et 160 millions de passagers par an, ce qui correspondrait à un quasi-doublement de sa fréquentation actuelle. Il s'agit là d'un atout majeur pour attirer le trafic aérien en correspondance, car plusieurs autres grands aéroports européens font aujourd'hui face à un phénomène de saturation. C'est le cas notamment de l'aéroport de Heathrow, à Londres, et de l'aéroport de Francfort. À l'issue de cette brève présentation, nous pouvons tous nous accorder sur ce point que la privatisation d'ADP se fasse ou non, l'État devra impérativement être en mesure d'assurer un contrôle étroit sur cette entreprise ... C'est indispensable ! ... et sur les infrastructures critiques dont elle assure la gestion. Il s'agit là ni plus ni moins d'un enjeu de souveraineté. Quelques mots sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous attendions avec impatience cet article 44 : le voici

ADP verse un peu moins de 180 millions d'euros de dividendes et vous attendez de ce fonds qu'il rapporte environ 200 millions d'euros. On sait

je vous confie mon PEL ! Je voudrais vraiment que vous nous répondiez sur cette question parce que cet argument économique ne tient absolument pas la route. La je vous remercie vous nous proposez aujourd'hui de privatiser des actifs hautement sensibles, des actifs hautement stratégiques. Après la privatisation ratée de l'aéroport de Toulouse, vous faites un peu plus fort en nous proposant de privatiser ADP,

qu'on fasse des erreurs, c'est une chose- et tout le monde en a fait -, mais qu'on les perpétue, c'en est une autre, c'est autrement plus grave ! On s'apprête, avec cet article,

à des mannes financières ou à des profits purement financiers ? ADP est un aménageur national et international, c'est la porte de la France sur le monde,

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en ce qui me concerne, je suis résolument opposé à la privatisation d'ADP, comme je l'ai été à celle de la Française des jeux. Ce n'est pas un principe ou un dogme, puisque j'ai soutenu la privatisation d'Engie. Donc, pas de procès d'intention Je suis opposé au transfert d'un monopole d'État à un groupe privé. L'expérience catastrophique du transfert des autoroutes n'a fait que me conforter. Voyez les conclusions de la commission d'enquête du Sénat ADP verse à l'État des dividendes, et il est donc étonnant de vendre au privé ce qui rapporte à l'État. Sur le plan international, avec les ports, ce sont les principales portes d'entrée, c'est notre frontière. également un sentiment de malaise, entre la privatisation d'ADP et l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, qui fut pour le Grand Ouest une faute impardonnable.

C'est une clientèle totalement captive, qui fait tourner l'ensemble de la plateforme commerciale, grâce aux investissements de l'État, donc grâce aux investissements des Français. L'aéroport, c'est un tout, et c'est la raison pour laquelle il faut revoir le principe des deux caisses : cela permettra à ADP de fixer des redevances d'un montant beaucoup plus raisonnable pour nos compagnies aériennes.

Monsieur le ministre, nous sommes favorables à la création de ce fonds, mais en l'alimentant avec les économies de fonctionnement sur la dépense publique et non en vendant les actifs rentables de l'État.

nous abordons la série d'articles qui concernent la privatisation d'Aéroports de Paris. Permettez-moi de vous rappeler un précédent fâcheux, celui de la privatisation de l'aéroport de Toulouse. L'État avait alors vendu 49,99 % du capital de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse à Casil Europe. de commerce et d'industrie locale ne possèdent ensemble que 40 % et l'État 10,01 %. La présence des collectivités locales au capital n'a pas empêché les dérives. En 2017, ces actionnaires publics locaux ont tenté en vain de s'opposer au groupe chinois et à sa volonté de maximiser le versement des dividendes au détriment des investissements. Au début de l'année dernière, l'État, fort heureusement, a décidé de conserver le peu de capital qu'il possédait encore et sur lequel le groupe Casil Europe avait pris une option. Un rapport de la Cour des comptes avait d'ailleurs critiqué en novembre 2018 un acquéreur dont le profil soulève des inquiétudes quant à son manque d'expérience en matière de gestion aéroportuaire, son manque de transparence financière et ses liens avec la puissance publique chinoise. Finalement, les investisseurs chinois ont récemment décidé de revendre leur participation, mais les craintes de la Cour des comptes demeurent. Cette privatisation reste inaboutie, la situation, ambiguë et instable. Cette revente n'efface pas le risque de voir une entreprise au capital majoritairement public, mais dont le contrôle est assuré par un actionnaire privé. Est-ce le sort qui attend Aéroports de Paris, entreprise capitale à la fois pour notre économie et pour notre souveraineté nationale ? Monsieur le ministre, je voudrais vous rappeler les propos que vous avez tenus au Sénat le 8 mars 2018 devant la mission d'information sur l'avenir d'Alstom : « L'État actionnaire doit être présent dans des secteurs stratégiques où notre souveraineté est en jeu. [ ...] Chacun peut comprendre que dans ces secteurs stratégiques, l'État a une place à occuper. Enfin, le rôle de l'État actionnaire, c'est aussi de garder une capacité d'intervention lorsque des des déséquilibres sont manifestes et qu'il faut réagir face à des décisions du secteur privé qui seraient injustes ou iniques. » Aussi, monsieur le ministre, permettez-moi d'exprimer ma totale incompréhension : entre vos propos que je viens de citer et la volonté du Gouvernement de privatiser ADP, il y a une véritable contradiction. Pourquoi ne considérez-vous pas ADP comme une entreprise stratégique ? Aux États-Unis, la quasi-totalité des aéroports sont publics et il est particulièrement inquiétant que l'État se désengage d'ADP. Céder ce groupe à des intérêts privés serait une vraie perte pour notre économie : en France aussi, la puissance publique doit rester majoritaire dans de telles infrastructures.

Là, privatiser un monopole, c'est aberrant, c'est créer une inégalité et c'est produire ce capitalisme des inégalités

il vous faut 9 milliards d'euros pour l'extension de l'exonération de la taxe d'habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés ; il vous faut 11 milliards d'euros pour financer les mesures d'urgence économiques et sociales que nous avons adoptées dans les conditions que vous savez, mes chers collègues, à la fin du mois de décembre. Donc, il vous faut beaucoup de, monsieur le ministre, et ces privatisations, qui s'inscrivent dans une période de croissance extrêmement fragile- les chiffres de l'INSEE nous le démontrent -sont finalement une mauvaise illustration d'une gestion aléatoire de notre pays. Vous voulez d'abord renflouer les caisses asséchées de l'État, mais c'est du, comme l'ont bien

pour continuer d'enregistrer des bénéfices, ces entreprises florissantes. S'il n'y avait pas d'exemple dans le passé, on pourrait vous excuser et croire à l'inexpérience, mais il y a l'exemple rappelé à plusieurs reprises de ces sociétés autoroutières, lesquelles se positionnent aujourd'hui sur les aéroports pour anticiper la future perte de leurs concessions. Mais l'État est-il là pour pallier la perte de ces concessions, alors que beaucoup contestent aujourd'hui la pertinence de ces privatisations ? Est-on obligé, monsieur le ministre, de faire une erreur pour pallier la fin d'une autre erreur ? ADP, l'exemple de l'aéroport de Toulouse, qu'a rappelé notre collègue Viviane Artigalas, montre bien que le choix a été aussi aléatoire. Monsieur le ministre, les infrastructures structurantes de notre pays sont des outils stratégiques que la collectivité publique doit continuer d'administrer

pas une opposition de principe, mais il soulève de réels problèmes. Monsieur le ministre, tout cela devrait vous alerter. Vous ne pouvez pas avoir raison tout le temps et contre tout le monde. Écoutez pour une fois le Sénat, ne bradez pas notre patrimoine, le patrimoine des Français.

avancés, il n'est pas inutile d'en ajouter quelques autres. Moi, je ne crois absolument pas à l'alibi de la nécessité de vendre les bijoux de la République pour constituer un pseudo-fonds d'innovation. Ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup : il serait nécessaire de vendre des entreprises ou des infrastructures pour, soi-disant, préparer l'avenir ! Toujours le même discours

%. On se prive donc de recettes à moyen et long termes pour du à court terme, lequel n'a jamais soutenu ni l'innovation ni la croissance ! Et que l'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas trouver de l'argent pour l'innovation en France.

risques d'une privatisation sont connus : gestion à l'économie, hausse des taxes aéroportuaires, pression sur les pouvoirs publics pour réduire les exigences environnementales et autoriser davantage de vols de nuit.

l'avons eu sur les nationalisations et, à de nombreuses reprises, sur les privatisations. Laissez-moi vous rappeler deux ou trois faits de notre récente politique économique

l'ont dit, les arguments sur le financement de l'innovation ne tiennent pas, puisque les dividendes suffiraient, suffiront, je l'espère, à financer l'innovation dans notre pays. Non, l'unique but de ces privatisations, et de celle-là, c'est effectivement un désendettement de façade relativement artificiel de notre pays, pour ne pas continuer à frôler la barre des 100 % du PIB. Là est l'unique souci. Mais pour ce faire, faut-il vendre, cela a été dit, un actif stratégique ? Monsieur le ministre, nous débattons aujourd'hui de ce texte au Sénat, avant qu'il revienne à l'Assemblée nationale. Mais, je vous le dis, les Français ne sont pas d'accord avec cette privatisation. Les Français ne sont pas d'accord avec ces privatisations, car ils en ont vu, s'agissant des autoroutes, les conséquences. Ils voient aujourd'hui ce que nous faisons, et ils ne sont pas d'accord. Vous n'avez pas le droit le droit juridique, vous l'avez -, pas plus que le droit moral de nous soumettre aujourd'hui cette question. Monsieur le ministre, le Président Macron cherche une question pour un référendum. Eh bien, suggérez-lui celle-ci

Qu'attendent les passagers ? Ils attendent de nous que nous soyons capables de promouvoir un système aéroportuaire efficace permettant la connectivité, la qualité de service et des prix raisonnables. Qu'attendent les compagnies qui nous regardent ? Que le Sénat soit capable aussi d'apporter sa pierre pour un développement du transport aérien. La France est une grande nation aérienne, elle a besoin de conforter cette place. On peut le faire en privatisant, on pourrait le faire en restant en gestion publique, mais maintenant que le Gouvernement a engagé ce processus, maintenant que l'Assemblée nationale s'est mise dans ses pas, il s'agit de voir dans quelles conditions nous pouvons agir et ce que le Sénat peut apporter pour contraindre le dispositif, pour le renforcer et y faire figurer un certain nombre de précautions qui seront utiles pour garantir les intérêts de l'État et ceux du transport aérien. Je crois que c'est cela, pour nous, faire oeuvre de législateur.

de M. Montebourg. Le texte était d'abord un texte de M. Montebourg ! Lyon et Nice, qui sont des projets de M. Macron, se sont bien déroulés et ne posent pas de problème particulier aujourd'hui. Deuxième point, le secteur aéroportuaire est quand même ouvert à la concurrence, on fait mine de l'oublier. Les passagers choisissent

Sénat dans ce texte. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article. J'aurai l'occasion de revenir sur les raisons de notre opposition à cette privatisation lors de l'examen des amendements. Pour l'heure, je souhaiterais, mes chers collègues, revenir sur un événement tout récent

Aujourd'hui, il est largement contesté par la population et nombre d'élus, qui souhaitent voir priorisés les transports du quotidien, notamment la ligne B du RER. Alors que Mme la ministre chargée des transports, sous la houlette de M. le préfet de la région d'Ile-de-France, a lancé une grande concertation sur l'opportunité de la réalisation de cette infrastructure, et que celle-ci n'est pas terminée, les faits témoignent d'une volonté d'avancer à marche forcée et en catimini. La coïncidence du calendrier nous interpelle, tout comme le comportement du Gouvernement à l'égard des élus et des populations locales dans ce dossier. Personne ne peut ignorer le lien entre le Charles-de-Gaulle Express et la privatisation d'ADP. D'un côté, l'État brade aux intérêts privés Aéroports de Paris et, de l'autre, il s'engage à hauteur de 1,7 milliard d'euros, dans le cadre du projet Charles-de-Gaulle Express, pour équiper gratuitement le futur repreneur de l'aéroport de Roissy : un État schizophrène qui organise donc sa propre impuissance en bradant ses intérêts. Il s'agit, pour nous, mais pas seulement pour nous, d'un coup de force inacceptable, et ce à plusieurs titres.

pour la révision des lignes. Inacceptable, ensuite, pour les élus et les associations engagés dans le processus de concertation. Inacceptable, enfin, pour l'ensemble de nos concitoyens, car ceux-ci devront, par leurs impôts, financer un équipement qui bénéficiera exclusivement à une société privatisée. Donc, en toute cohérence, nous continuons à demander la suspension du projet Charles-de-Gaulle Express, et nous portons dans cet hémicycle la voix de la préservation des intérêts de notre pays en refusant la privatisation d'ADP.

Aéroports de Paris, la Française des jeux et ENGIE. Je veux dire ici mon opposition frontale à ces privatisations et, d'abord, à celle d'Aéroports de Paris. Le premier argument avancé, le financement du fonds consacré à l'innovation, a déjà été démonté dans l'intervention précédente, au regard des dividendes perçus chaque année par l'État. les privatisations amélioreront la gestion de ces entreprises en leur appliquant les bonnes pratiques des groupes privés, n'est qu'une pétition de principe teintée d'idéologie sans aucun fondement. Dans le cas d'un monopole comme ADP, le confier au secteur privé revient à lui remettre une forme de rente que rien ne justifie, à l'image de la privatisation des autoroutes, dont pâtissent les Français. de la dette publique, ne convainc pas davantage. ADP possède un caractère stratégique incontestable. Première porte d'entrée en France, il joue un rôle touristique majeur, mais aussi un rôle clé en matière sécuritaire. Il a réalisé, l'an passé, un chiffre d'affaires accueilli plus de 100 millions de passagers. Les locations d'espaces aux grandes marques de luxe et de restauration représentent désormais un tiers du chiffre d'affaires. Pourquoi, mes chers collègues, priver l'action publique et l'intérêt général d'un avenir qui est annoncé prometteur ? Une folie ultralibérale en matière aéroportuaire conduit, mes chers collègues, à une aberration économique, à une erreur stratégique, à une faute politique politique majeure, alors que, dans le même temps- cela a déjà été évoqué -, la Cour des comptes, dans son rapport d'octobre 2018, relève que l'arrivée d'acteurs privés ne s'est pas accompagnée d'inflexions majeures en matière de gestion et d'orientation stratégique des trois aéroports concernés : Toulouse, Lyon et Nice. je vous remercie vous ne pouvez plus ignorer que cette question de la privatisation d'Aéroports de Paris occupe désormais une place particulière dans nos débats. Au demeurant, je trouve que cette question, qui vient au débotté dans ce projet de loi fourre-tout, aurait mérité un texte à part. part. De nombreuses critiques mettent en avant le risque de bradage d'un emblème national et d'une infrastructure stratégique au profit du secteur privé. Vous affirmez, de votre côté, votre volonté de voir l'intérêt public préservé, mais cela ne suffit pas à nous rassurer, puisque nous sommes tous conscients ici des risques que cette privatisation, d'un monopole de surcroît, représente. Le parallèle avec la privatisation des autoroutes a été fait à de nombreuses reprises ici, notamment au regard du principal intéressé, pour le rachat d'ADP. Il y a Il y a bien un risque, effectivement, qu'un groupe, déjà actionnaire à hauteur de 8 %, détienne alors un monopole à la fois sur les autoroutes et sur les aéroports, deux secteurs stratégiques indispensables au bon fonctionnement de notre pays. Je dois vous le dire, monsieur le ministre, vos propos à la fois sur le cahier des charges, les redevances, les investissements, le statut des personnels ou encore le contrôle des frontières, ne sont pas de nature à nous rassurer. Enfin, le précédent fâcheux de la privatisation de l'aéroport de Toulouse, décidé en 2015 par le gouvernement d'alors, devrait nous alerter un peu plus sur les risques d'une telle décision. Les investisseurs chinois qui ont racheté en 2015 l'aéroport de Toulouse cherchent aujourd'hui à le revendre, en faisant une confortable plus-value de 200 millions d'euros en quatre ans seulement. Encore une fois, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas minimiser ou évacuer le risque réel que représente cette privatisation de nos infrastructures stratégiques en les laissant à la merci des actionnaires, et, plus encore, des pratiques douteuses qu'a révélées dernièrement la Cour des comptes lors d'un précédent rapport. je ne voterai pas cette privatisation, et donc je voterai les amendements tendant à sa suppression, car je ne peux pas, monsieur le ministre, vous suivre dans cette voie qui nous amène assurément dans une zone de turbulences dont l'issue serait grave pour notre pays.

Troisièmement, dans le pays le plus libéral au monde, les États-Unis, la souveraineté existe et les aéroports restent dans le domaine public. Je dirai que je suis libéral parce que, vous l'avez dit vous-même, l'État défend mal ses intérêts. Dans ce dossier, ce constat est particulièrement vrai, et la démonstration

Malgré ce déséquilibre, qui semble flagrant sur la dévalorisation, on ne parle qu'à situation constante, c'est-à-dire aujourd'hui et pas dans soixante-dix ans. Or M. le rapporteur nous dit que le trafic va exploser dans les prochaines décennies. Et vous n'avez même pas prévu de clause de

Permettez-moi de vous citer, monsieur le ministre : « Nous avons défini un cahier des charges strict. Vous avez manifesté une inquiétude légitime au sujet des redevances. Les deux redevances seront négociées tous les ans et l'État aura le dernier mot sur leur niveau. » Vous avez même ajouté : « Le cahier des charges permet de renforcer le contrôle de l'État par rapport à la situation précédente Monsieur le ministre, il nous faut plus que de simples paroles pour nous convaincre lorsque l'on s'apprête à privatiser l'un des premiers aéroports d'Europe qui, de plus, est l'employeur de 6 400 salariés. Nous ne pouvons débattre sérieusement et voter cet article sans un document écrit. Vous comprenez, nous n'avons pas confiance. Quels sont les critères choisis pour ce cahier des charges ? Quelles sont les obligations de service public et de sécurité ? Vous nous dites que le cahier des charges intégrera les amendements sur le statut des personnels et de l'emploi et que les intérêts de l'État seront évalués plus régulièrement. Mais quelles garanties avons-nous réellement sur le maintien de ces dispositions et sur les autres critères de ce cahier des charges ? Aussi, je vous pose une question toute simple, monsieur le ministre : où est le cahier des charges ? Nous devons disposer d'une information complète pour nous prononcer, sans quoi nous vous donnons carte blanche pour liquider nos services publics de qualité au premier investisseur étranger venu. Ce que nous vous demandons est pourtant simple. J'ai ici avec moi l'actuel cahier des charges d'Aéroports de Paris qui date de 2005. Nous Nous voudrions savoir ce qui va changer dans le futur cahier des charges pour pouvoir nous prononcer. J'attends donc votre réponse, monsieur le ministre de l'économie et des finances. La parole

à un, à deux, voire à trois grands groupes dans notre pays, l'ensemble des déplacements stratégiques nationaux et internationaux. En réalité, la problématique que vous posez sur la maîtrise ou non du monopole, vous vous en dégagez en renvoyant vers pour ne pas les citer. Vous nous avez dit ici, la semaine dernière, que l'enjeu de la privatisation d'Aéroports de Paris, c'était la gestion des boutiques. Mais sérieusement, monsieur le ministre, l'enjeu de la privatisation d'Aéroports de Paris et des conséquences stratégiques, y compris en termes d'aménagement du territoire, sur l'ensemble de l'Île-de-France et bien au-delà, peut-il se résumer simplement à savoir qui gérera ou pas demain, et selon quel niveau de concurrence, les boutiques d'Aéroports de Paris, sauf à se dire que ces boutiques doivent devenir demain des arènes de combat pour certains rappeurs en manque de sensations

mais des entreprises stratégiques en termes d'emplois et de développement, dans les années qui viennent, pour notre pays. Je finirai sur une remarque, monsieur Yung. Vous avez cité plusieurs exemples de privatisation

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous pensons que la privatisation d'ADP est contraire à la Constitution.

vous le dites dans le grand débat national aux Françaises et aux Français ? Et lorsque les entreprises deviennent trop puissantes, la séparation du politique et de l'économique disparaît. Notre Constitution, en son préambule, avait prévu ce risque, et posé la nécessité d'un pouvoir de contrôle et de police économique de ces biens essentiels. Vous nous avez dit, monsieur le ministre, au commencement de l'examen de cette loi, qu'ADP, ce sont des hôtels et des boutiques de luxe, que l'État n'a pas à gérer. Pour nous, ADP est un monopole naturel, un service public national qui devrait, à ce titre, échapper à la privatisation. Il faut le justifier. C'est pourquoi de nombreux juristes, et pas des moindres, s'élèvent aujourd'hui aussi contre cette privatisation. Le Conseil d'État soutient que le préambule de la Constitution de 1946 ne peut être invoqué contre un projet de loi, car tout en reconnaissant le caractère de service public d'ADP, il énonce que sa situation géographique exclurait qu'il puisse s'agir d'un service public national, puisque la mission de service public confiée à ADP ne s'exercerait que sur la seule région d'Île-de-France. Il ne serait pas non plus un monopole de fait.

et exclut la quasi-totalité des services publics existants. Or ADP, c'est treize aéroports, des participations dans de nombreux aéroports à l'étranger, des filiales avec des activités d'ingénierie, de gestion et de développement aéroportuaire. Le seul aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle devrait avoir à gérer un flux de 120 millions de passagers par an d'ici à 2023, date de mise en service du terminal 4, qui en ferait le premier aéroport européen. ADP joue un rôle considérable dans l'aménagement du territoire national, à la fois par son poids économique pour la région capitale, mais aussi par son utilité pour le transport interne à la France, aussi bien en métropole que dans le lien entre celle-ci et les départements et territoires d'outre-mer, comme le Sénat le rappelait déjà en 2005. ADP, c'est aussi un monopole de fait, puisque les secteurs d'activité sur lesquels la société détient une position exclusive ou prépondérante, occupent une place importante et non substituable dans l'économie nationale. De plus, ces secteurs d'activité représentent la majeure partie de son activité globale. Je vais vous le dire, monsieur le ministre, comme d'autres l'ont dit ici, même si j'aborde un aspect plus juridique, on est en train de faire un choix idéologique et politique, c'est d'avoir des lectures différentes de notre Constitution. Il faut

Allez-vous céder plus de 50,2 % en un bloc, en plusieurs blocs ? Va-t-il y avoir une OPA ? Comment seront choisis ceux qui vont éventuellement

Comment allons-nous protéger notre aéroport dans le temps d'une future possible OPA sur un secteur d'activité ouvert ? Nous avons donc là des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Alors, vous nous rassurez, en disant : « Nous maîtriserons la sécurité. Nous maîtriserons le contrôle des frontières. Nous maîtriserons toutes les compétences régaliennes. Nous maîtriserons le montant et la nature des investissements, ainsi que le devenir du foncier ».

Or sur ce sujet précisément, il y a une très grande convergence d'analyses, de diagnostics et de questions. En vérité, il y a une raison

Quand je regarde les outils destinés à mettre en oeuvre le fonds d'innovation stratégique, j'observe qu'une première enveloppe sera utilisée sous forme d'aides individuelles- subventions, avances remboursables ou prêts. Ce sont les outils des investissements d'avenir ! Je lis qu'une seconde enveloppe financera des programmes répondant à des défis à fort enjeu technologique l'intelligence artificielle, pour 100 millions d'euros par an, la nanoélectronique, pour 25 millions d'euros par an. Si je lis le projet annuel de performance du programme des investissements d'avenir pour l'année 2019, je constate qu'un certain nombre de fonds ont déjà été réorientés vers l'intelligence artificielle, d'où mes questions

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat est animé, et c'est tout à fait normal,

pour améliorer ce texte et renforcer les garanties accordées à nos compatriotes, dans le cadre de la cession des actifs de l'État dans Aéroports de Paris.

de sel. Madame Lienemann, il me semble que, lorsque M. Jospin était Premier ministre, vous ne défendiez pas avec autant d'ardeur le refus des privatisations également assez piquant de voir certains sénateurs Les Républicains- pas tous : certains posent des questions, d'autres sont plus péremptoires -dénoncer avec tant de vigueur les privatisations. Je leur rappellerai simplement une citation Il faut reprendre les privatisations et que l'État reprenne des capitaux immobilisés dans des entreprises commerciales où il a gardé des participations, qu'on récupère cet argent et qu'on investisse ». C'était François Fillon, c'était en 2016, et c'était son programme pour la présidentielle. Et ça s'est mal terminé

je tiens à dire très clairement à quoi sert cette opération. Elle a trois buts : le financement du fonds pour l'innovation de rupture, le désendettement de notre pays et la création

plutôt que des rendements instables et incertains. En 2008, les dividendes étaient de 110 millions d'euros. En 2010, ils sont tombés à 70 millions d'euros- ce qui représente 40 millions d'euros

Il ne me semble pas totalement absurde de confier la gestion des boutiques, des hôtels et du développement international d'Aéroports de Paris au secteur privé : c'est ma conviction.

: les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires français sont capables de faire mieux que les Américains, qu'il s'agisse de la qualité de service des aéroports ou de la valorisation des infrastructures aéroportuaires.

ne serait pas rentable, mieux vaudrait compter sur les recettes des dividendes, qui seraient régulières dans le temps, pour alimenter notre fonds pour l'innovation de rupture.

fait une comparaison avec les autoroutes. Mais comparaison n'est pas raison : ces deux opérations n'ont strictement rien à voir, pour des raisons fondamentales.

Une disposition législative, un renforcement de l'autorité indépendante : cela nous distingue totalement de l'opération relative aux autoroutes, et cela vous garantit le contrôle de l'État sur les tarifs aéroportuaires.

Le contrôle sera plus fort après la loi PACTE qu'il ne l'était avant ; les dispositions de caractère législatif

Paris. Ce cahier des charges est un élément absolument structurant des garanties apportées à Aéroport de Paris. Votre rapporteur a suggéré qu'il fasse désormais l'objet d'une clause de revoyure tous les dix ans.

Le contrat de régulation économique devenant une disposition législative ; le renforcement de l'autorité indépendante ; le cahier des charges, que nous mettons à votre disposition et que je suis prêt à voir réexaminer tous les dix ans

La conclusion que je tire de tous ces éléments que je tenais à porter à votre connaissance est la suivante : l'opération qui vous est proposée permet, au bout du compte, à l'État de récupérer cet actif stratégique ; elle se fait avec trois verrous sûrs que sont le renforcement de l'autorité indépendante,

Fabien Gay, je ne reviens pas sur votre PEL,

et, de l'autre côté, un fonds placé à 2,5 % qui garantit rentabilité et sécurité pour l'innovation de rupture. Monsieur Martial Bourquin, vous avez développé un argumentaire qui a été repris par beaucoup d'autres sénateurs sur le monopole d'État.

de cela. En la matière, c'est la meilleure garantie que je peux vous donner. Monsieur Olivier Jacquin, vous nous dites que nous faisons cela parce que nous avons besoin d'argent. Non, nous faisons un choix d'investissement.

Je préfère que l'on ne s'engage pas sur ce chemin, parce qu'il ne me semble pas que gestion des socialistes de 2012 à 2017 ait été un modèle de bonne gestion.

pour Emirates ou pour n'importe quelle autre compagnie du Moyen-Orient en privatisant ou pas Aéroports de Paris, la DGAC continuera à les accorder aux compagnies aériennes étrangères. Ne jouez pas avec les peurs des Français

ou, au contraire, essayer d'améliorer le texte qui est entré au Sénat. Je préfère cette seconde option et c'est avec cette attitude que je me présente à vous aujourd'hui et que je réponds à vos questions.

Monsieur Yves Daudigny, je ne reviens pas sur la comparaison entre les autoroutes et leurs péages et les aéroports, j'ai déjà fait valoir suffisamment d'arguments à ce sujet.

particulier d'inquiétude, sans compter que les opérations sur les aéroports de Toulouse, Lyon et Nice n'étaient pas entourées des mêmes garanties que celles que nous apportons aujourd'hui.

Je veux simplement vous assurer que, au titre du cahier des charges, que vous avez proposé de revoir tous les dix ans, il est prévu que toute modification de l'utilisation et de l'usage de ce foncier non encore bâti nécessite l'accord de l'État.

je conteste absolument le raccourci qu'elle a fait entre les privatisations et la montée du Front national. J'ai rarement entendu cet argument, c'est le mérite du débat parlementaire, mais je ne vois absolument aucun lien entre privatisations et montée du Front national. En revanche,

dans les technologies d'avenir et d'avoir un fonds de financement des innovations de rupture qui permette à nos industries d'être à la pointe des technologies qui créeront des emplois demain. Si vous voulez lutter contre la désindustrialisation, soutenez le fonds pour l'innovation de rupture et l'opération qui vous est soumise aujourd'hui

Ce n'est pas l'avis du Conseil d'État, lequel a estimé qu'Aéroports de Paris n'était pas un monopole naturel et n'avait pas vocation à être un service public national. Il y aura des recours, c'est légitime, et le Conseil constitutionnel tranchera, mais nous nous sommes fondés sur l'avis juridique du Conseil d'État, qui me semblait être le mieux placé en la matière.

Rien n'a été tranché sur les modalités de cette opération et j'attends de nos débats qu'ils permettent de nous éclairer sur ce que les parlementaires jugent le plus pertinent en matière de cession des actifs de l'État.

je suis ouvert à ce que la région Île-de-France soit représentée comme censeur au conseil d'administration d'Aéroports de Paris après l'opération. après l'opération. En résumé, et je terminerai par les trois dernières questions qui m'ont été posées, mais en rebondissant sur la question de Mme Primas, je vous propose donc que nous discutions des modalités de cession,

Monsieur Pierre Laurent, vous me dites que les arguments que j'ai avancés étaient trop légers, je pense vous avoir convaincu, juste avant le dîner, qu'ils pouvaient être un peu lourds quand c'était nécessaire ! Monsieur Claude Bérit-Débat, j'ai déjà répondu Madame Christine Lavarde, la question des investissements d'avenir est très importante. Nous manquons de fonds pour des recherches sur des technologies très pointues très sensibles sur lesquelles il faut investir, parfois pendant des années et des années à fonds perdus. Je pense, par exemple, un projet de financement, par ce fonds pour l'innovation de rupture, d'une étude sur le biais de sélection des algorithmes, qui est un sujet démocratique fondamental. Vous regardez votre iPhone et vous voyez des alertes de presse. Pourquoi telle information est-elle sélectionnée plutôt que telle autre ? Comment l'algorithme a-t-il choisi de vous faire parvenir telle information plutôt que telle autre ? Pourquoi tel relais d'opinion va-t-il arriver chez tel citoyen, plutôt que tel autre ? Nous le constatons à la faveur de la crise des « gilets jaunes

mais n'est rentable pour aucune entreprise. C'est pourquoi nous avons décidé de faire financer cela par le fonds pour l'innovation de rupture. Les programmes d'investissements d'avenir ne correspondent pas à ce type de recherches, qui sont plus pointues, plus difficiles, mais pas moins essentielles pour l'avenir de notre pays.

que cette cession d'actifs de l'État est l'occasion de redéfinir clairement les rôles respectifs de l'État et de l'entreprise dans notre société. Notre nation a besoin d'un État qui nous protège, qui investisse dans l'innovation, dans la technologie, dans la recherche. C'est également ce qui vous est proposé ici. dans cette opération.

que la seule personne qui n'ait pas pu s'exprimer jusqu'au bout fût notre rapporteur, qui a travaillé sur ce sujet et qui, au terme des deux minutes trente qui lui étaient allouées, a été contraint de reporter son explication. Beaucoup d'entre nous, qui ne connaissent pas le sujet parce qu'ils n'appartiennent pas à la commission, mais qui ont des idées assez arrêtées sur l'économie en général, sur les infrastructures, sur leur détention et leur propriété, auraient

Une bonne partie des membres du groupe socialiste et républicain s'est exprimée. Dans notre majorité sénatoriale, ceux qui ont des réserves sur ce projet ont pu les exprimer, c'est bien normal, mais celui qui porte notre message n'a pas pu s'exprimer et ce n'est pas tout à fait normal.

qui fait des bénéfices, qui investit et qui a beaucoup changé la donne des aéroports franciliens. Elle a beaucoup travaillé avec les collectivités, avec la région, avec les départements et a bénéficié de nombreux aménagements,

les critiques de cette privatisation émanent de l'ensemble des travées du Sénat, gauche et droite confondues. Si nous faisons ensemble

Ensuite, il a montré que nous vous proposons une opération originale, dans laquelle toutes les garanties d'encadrement par l'État sont apportées.

n'est pas de gérer à 73 % le développement international d'Aéroports de Paris, des boutiques ou des hôtels. Le rôle de l'État est de garantir la sécurité de nos frontières et d'investir dans l'avenir de nos enfants. si vous approuvez la cession des actifs de l'État dans Aéroports de Paris, vous permettrez à l'État de se concentrer sur ses missions essentielles, la protection des Français et l'investissement dans l'avenir de nos enfants, et vous laisserez à un opérateur privé, sous le contrôle étroit de l'État, le soin de développer nos infrastructures aéroportuaires

de débattre de la privatisation des aéroports, en particulier de Roissy-Charles-de-Gaulle, avec une telle perspective d'augmentation du trafic, alors même qu'une procédure de concertation vient juste de commencer pour la construction d'un quatrième

beaucoup attiré l'attention : les conséquences de la privatisation d'ADP pour notre compagnie nationale, Air France, lesquelles plaident pour la suppression de l'article 44. Pour que l'État puisse vendre ADP à un très bon prix, il faut qu'il puisse faire espérer au futur acquéreur privé des résultats en croissance. Pour cela, il faudrait qu'il dérégule les redevances aéroportuaires qu'il fixe aux compagnies aériennes et aux passagers. Or s'il acceptait d'augmenter ces taxes, Air France pourrait en souffrir, puisque quasiment tout son trafic passe par les aéroports parisiens. Ainsi, l'alternative est simple soit l'État continue à réguler l'augmentation des redevances, au risque de faire une mauvaise opération en vendant à bas prix ; soit il lâche du lest, mais ce sont les passagers et Air France qui en souffriront. De plus, lors de son audition par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, M. Benjamin Smith, nommé directeur général d'Air France en août

identiques de suppression, car je suis contre la privatisation d'ADP. À mon sens, on ne doit pas permettre à une entreprise privée d'exercer un monopole sur une infrastructure stratégique. infrastructure stratégique. Les infrastructures stratégiques, comme les ports maritimes, certains aérodromes civils et les sites de production, de réseau et de distribution d'énergie électrique, doivent demeurer incessibles. En effet, il paraît logique et responsable de garder la main sur ce qui est d'un intérêt national supérieur, car c'est une question de souveraineté. C'est un principe de base, un principe fort, un principe républicain : la finance ne peut pas prévaloir sur tout ! Permettez-moi de souligner une

ce qui m'a été répondu : « L'exonération de péage pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération constitue une rupture d'égalité des usagers devant le péage. Il s'agit, pour les sociétés concessionnaires, d'une charge nouvelle qui leur est imposée et pour laquelle elles ne pourraient être compensées par une hausse des tarifs de péage. [ ...] Les sociétés concessionnaires pourraient donc se prévaloir d'un préjudice devant le juge du contrat, comme elles l'ont déjà indiqué à l'État.

1,4 % du PIB national et 8 % de l'emploi salarié francilien, emplois directs et induits confondus. L'augmentation du trafic aérien et du nombre de passagers devrait impliquer un renforcement des métiers d'ADP. Or, aujourd'hui, les salariés et leurs syndicats dénoncent

au service de l'innovation. Même si l'objectif est louable, on est dans une logique d'opportunité. Il aurait été préférable de débattre de la vision stratégique

ceux de Hong Kong, Séoul, Singapour, Dubaï et Amsterdam-Schiphol, sont sous gestion publique. Preuve que, dans un monde en pleine évolution où le transport aérien va exploser dans les années qui viennent, une prise en main de la part de l'État est

mais si vous voulez vraiment que le Sénat joue son rôle, il faut aller au fond des choses et permettre la navette. Concernant le fond, vous nous expliquez que cette privatisation vise à préparer l'avenir parce qu'il faut investir. Vous seriez plus crédible, permettez-moi de le dire aussi simplement, si le budget de 2019 s'était traduit par une moindre dépense publique et une moindre augmentation de la dette. Enfin, vous nous expliquez que cette privatisation revient à voir très loin.

en faveur du droit d'entreprendre, contre l'intérêt général. Notre culture administrative n'est pas portée sur le contrôle, comme peuvent l'être les économies libérales de type anglo-saxon, qui se dotent véritablement

de 1 milliard d'euros, si ma lecture est correcte, sera versée aux actuels actionnaires minoritaires, parmi lesquels le groupe Vinci, de la société ADP. Cette indemnité d'expropriation est non pas préalable à une renationalisation, qui interviendra dans soixante-dix ans et que connaîtront peut-être nos enfants ou petits-enfants, mais en partie concomitante à la privatisation,